Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris la mort, samedi dernier, du brigadier Alexandre Martin, du 54 régiment d'artillerie d'Hyères. Alexandre Martin a succombé à ses blessures à la suite de l'attaque du camp français de Gao, au cours de laquelle plusieurs autres de ses frères d'armes, nos soldats, ont également été touchés. Au nom du Sénat tout entier, je veux saluer le courage de ce soldat, mort pour la France en luttant contre le terrorisme djihadiste au Sahel, et exprimer notre solidarité envers les blessés. En notre nom à tous, je veux assurer sa famille et ses frères d'armes de notre profonde compassion et leur présenter nos pensées et nos condoléances attristées. demande d'observer un court moment de recueillement en hommage à Alexandre Martin, qui a servi la France avec honneur et dévouement.

J'appelle chacun d'entre vous à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles du Sénat : le respect, qu'il s'agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps de parole.

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, et porte sur la situation aux frontières entre la Russie et l'Ukraine. Monsieur le ministre, le conflit russo-ukrainien semble s'aggraver de jour en jour et les tensions qu'il provoque entre les Russes et les Occidentaux deviennent de plus en plus préoccupantes. Hier encore, la Russie a effectué une série de manoeuvres militaires, impliquant 6 000 hommes, des avions de chasse et des bombardiers, le long de sa frontière sud avec l'Ukraine et Ces opérations interviennent après le déploiement de chars et de 100 000 soldats à la frontière ukrainienne, faisant craindre une possible invasion. Dans le même temps, l'Ukraine est également touchée par des cyberattaques ciblant notamment plusieurs sites gouvernementaux. l'Atlantique Nord) ont, pour leur part, placé des forces en alerte et envoyé des navires et des avions de combat pour renforcer la défense en Europe de l'Est. Réunis en visioconférence ce lundi, les dirigeants des États-Unis, des instances européennes, de l'OTAN et de plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne, ont réaffirmé leur soutien sans réserve à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ils ont évoqué des sanctions très lourdes à l'encontre de la Russie en cas d'agression contre ce pays. Parallèlement, des efforts diplomatiques, auxquels la France prend toute sa part,

a, quant à elle, pris l'initiative de relancer les rencontres et les discussions dans le format Normandie. Dans ce contexte, monsieur le ministre, comment la France compte-t-elle agir pour élaborer une position unique et forte

je ne vous cacherai pas que la situation est sous très grave tension. Comme l'a dit le Président de la République hier aux côtés du Chancelier allemand, la Russie se comporte comme une puissance de déséquilibre et il ne tient qu'à elle de devenir un acteur de désescalade. Nous sommes totalement mobilisés, avec nos partenaires européens, avec nos partenaires américains, pour enrayer la dynamique de l'escalade- il faut appeler les choses par leur nom.

Les entretiens que j'ai eus, avec le secrétaire d'État Blinken avant-hier, avec le secrétaire général de l'OTAN hier, montrent la force de cette unité autour de trois priorités. D'abord, des sanctions massives seront imposées à la Russie si elle porte une nouvelle atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous y travaillons. Ensuite, il faut tout faire pour que le dialogue avec la Russie se poursuive, afin de contribuer à la désescalade. Des discussions dans le format Normandie ont lieu aujourd'hui même à Paris.

de résilience européenne, mais aussi de contribution au dialogue. La présidence française est totalement mobilisée pour ces initiatives. Je me rendrai moi-même à Kiev dans quelques

sur votre perception de l'état de l'école, alors que le contexte de crise sanitaire affecte considérablement son fonctionnement depuis deux ans. Même si le ministre de l'éducation nationale défend ardemment ses réformes, son échec à la tête du ministère est patent. La réforme du lycée est ratée. Alors que son objectif était de casser l'effet filière, elle a accru les inégalités sociales et territoriales. Au collège, la diminution constante du nombre de postes pour privilégier les heures supplémentaires a abouti à un manque considérable d'effectifs, avec des remplacements non assurés, en particulier dans la période de crise sanitaire que nous vivons depuis deux ans. ans. À l'école élémentaire, la grande réforme du quinquennat, le dédoublement des classes de CP et de CE1 en zone prioritaire, produit des résultats classés par les chercheurs dans le bas de la fourchette. Cette réforme étant très consommatrice de postes, vous avez ponctionné des moyens sur un dispositif, appelé « Plus de maîtres que de classes », qui donnait pourtant entière satisfaction aux enseignants. enseignants. Bien que les textes prévoient toujours une semaine scolaire de neuf demi-journées, la quasi-totalité des écoles de ce pays fonctionne par dérogation sur quatre journées, un rythme dont on connaît la nocivité pour les enfants, mais qui satisfait nombre de lobbies périphériques à l'école. Enfin, rien n'a été fait pour revaloriser sérieusement les carrières et les formations des enseignants. Le métier n'est plus attractif et nous courons à la catastrophe pour les recrutements. Par ailleurs, la gestion de la crise sanitaire depuis deux ans est jugée erratique, irréaliste et inopérante par les enseignants, qui vous crient tous les jours leur souffrance. Madame la secrétaire d'État, comment le Gouvernement compte-t-il agir pour rétablir la confiance dans et autour de l'institution scolaire ? La parole est à Mme la secrétaire d'État

parmi les préoccupations majeures de nos concitoyens figure l'égal accès à des soins abordables et de qualité, dans tous les territoires, quelle que soit la situation matérielle d'un malade. Il n'est pas acceptable que nos concitoyens les plus précaires soient contraints de renoncer à des soins, surtout dans la situation sanitaire la mise en place depuis le 1 janvier d'un forfait patient urgences de 19,61 euros risque d'éloigner davantage des personnes déjà fragiles de l'accès aux soins, car elles ne pourront pas avancer les frais. près de 3 millions de personnes sont dépourvues de complémentaire santé et sont susceptibles de reporter des soins, ou d'y renoncer. Le recours aux urgences est aujourd'hui le seul moyen d'accéder à une prise en charge rapide dans les zones sous-dotées en médecins généralistes, en milieu rural comme urbain. Plus largement, c'est encore une fois la question du maillage du service public de la santé qui nous préoccupe. Le Président de la République l'a souligné hier dans la Creuse : le manque de médecins disponibles engendre une situation très critique, voire profondément inquiétante dans de nombreux territoires ruraux. Entre 6 et 8 millions de personnes vivent aujourd'hui dans un désert médical, où ni la médecine de ville ni des établissements de santé ne sont facilement accessibles. Il y aurait pourtant beaucoup à faire pour mieux articuler l'hôpital avec la médecine de ville.

d'attractivité économique : tous ces facteurs s'entre-alimentent constamment, créant une spirale négative qui paraît ne pas avoir de fin. Tous, nous sommes attachés au principe de l'égal accès au service public de la santé. santé. Comment comptez-vous renforcer les politiques publiques concourant à ce principe fondamental de notre République ? La parole est à M. le Premier ministre.

D'après la Cour des comptes, la France n'était pas préparée à faire face à la covid en ce siècle pourtant annoncé comme celui des pandémies. Pendant la crise, votre gouvernement, comme tous ceux qui l'ont précédé, a poursuivi les restructurations et les fermetures de centres hospitaliers. Selon la Drees, 25 établissements ont fermé en 2020. Les fermetures définitives de lits se multiplient, fermetures provisoires, par manque de personnel. Plus les mois passent et plus la situation devient critique. Selon le syndicat des infirmiers, 7 500 postes d'infirmiers étaient vacants en juin 2020

une initiative irrespectueuse envers les fonctionnaires hospitaliers en place, qui luttent depuis deux ans et qui voient cette pratique s'ajouter à l'intérim mercenaire. Quelle fuite en avant ! est de constater que, faute d'un changement radical du système de santé, le choc d'attractivité n'a pas eu lieu après le Ségur. Cette semaine, une nouvelle mobilisation des professionnels est prévue. Que compte faire le Gouvernement pour prendre enfin la mesure de la situation et stopper l'hémorragie de personnel ?

sont bien réelles, et elles ne sont pas nouvelles. Il est vrai qu'elles ont été amplifiées par la cinquième vague épidémique, avec le double impact des variants delta et omicron,

C'est désormais une certitude : l'inflation fait de nouveau partie du paysage économique. Elle s'établit à 5 % dans la zone euro, bien au-delà des prévisions des économistes. Heureusement, le choc est plus modéré en France. La question ne porte pas sur les causes de cette inflation. Personne ne remet en cause le « quoi qu'il en coûte ». Nos impôts ! Du moins, personne ne l'a contesté au plus fort de la crise, quand notre pays mobilisait ses forces pour lutter contre le virus. La question porte sur les conséquences, à court terme comme à long terme, de cette inflation. À court terme, le Gouvernement a mis en place des dispositifs d'urgence, qui ont largement atténué ses effets. Je ne veux pas relancer ces débats, que nous avons déjà eus ici. Ma question porte sur les conséquences à long terme de l'inflation. Parmi les scénarii possibles, celui d'un relèvement des taux d'intérêt inquiète. Ce risque n'a jamais paru aussi élevé. Aux États-Unis, le patron de la Banque fédérale a reconnu que l'inflation n'avait rien de transitoire. Il laisse entendre qu'il pourrait relever les taux pour éviter une crise sociale. En Allemagne, le rendement des obligations d'État à dix ans est repassé au-dessus de zéro, une première depuis 2019. Il est hautement improbable que la France soit épargnée. Face à cette hypothèse, notre pays a deux atouts : la croissance la plus forte et l'inflation la plus faible de toute la zone euro. Mais, madame la ministre, il a une faiblesse : sa dette publique. Le gouverneur de la Banque de France a rappelé hier que le taux d'entêtement actuel n'est pas soutenable à long terme. Ma question est donc simple, madame la ministre : comment évaluez-vous le risque de relèvement des taux d'intérêt ? Pouvez-vous nous rassurer sur la capacité de la France à rembourser sa dette ?

vous le signalez dans votre introduction, la France a deux atouts : la croissance la plus forte et l'inflation la plus faible

Ces mesures, utiles, laissent cependant sur le rebord de la route de nombreuses entreprises pénalisées à cause des effets de seuil ou des conditions d'éligibilité trop restrictives. Chaque semaine, je suis interpellée sur le terrain par des chefs d'entreprise exaspérés par ce qu'ils considèrent comme une usine à gaz. C'est le cas d'un restaurateur en grande difficulté financière, mais qui ne peut pas bénéficier ne peut pas bénéficier du dispositif Coûts fixes, car se situant juste en dessous des 50 % de chiffre d'affaires perdus ; ou encore d'un traiteur, exclu lui aussi du dispositif, bien qu'ayant perdu deux tiers de son chiffre d'affaires, mais avec un excédent brut d'exploitation positif parce qu'il a été contraint de réduire ses achats et son personnel en décembre. décembre. Vous comprendrez aisément l'exaspération et le sentiment d'injustice que peuvent ressentir ces professionnels. Ils ne s'expliquent pas pourquoi le « quoi qu'il en coûte » ne ruisselle pas jusqu'à eux. Quelles solutions concrètes pouvez-vous leur apporter alors qu'ils s'inquiètent un peu plus chaque jour pour leur avenir et leur survie ?

Madame la présidente,

Des usagers, des personnels et des responsables d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux viennent dénoncer les incohérences de la mise en oeuvre du Ségur de la santé.

vous avez annoncé le 8 novembre dernier qu'une conférence sur les métiers de l'accompagnement social et médico-social se tiendrait avant le 15 janvier. Nous sommes le 26 janvier, et il ne s'est rien passé. Qu'en est-il ?

depuis plusieurs mois par le Gouvernement pour soutenir les professionnels de santé et du soin dans le cadre du Ségur de la santé, après dix ans de sous-investissements. Le Ségur est de loin le plus important plan de soutien à notre système jamais engagé par une majorité présidentielle.

médico-techniques et de la rééducation depuis le mois d'octobre 2021. Les personnels médicaux ne sont pas en reste. Nous avons fusionné les premiers échelons de rémunération et amélioré leur fin de carrière avec des nouveaux échelons. Nous avons mis en place des primes managériales et revalorisé l'indemnité d'engagement de service public exclusif. Surtout, contrairement à l'idée selon laquelle il y aurait des « oubliés du Ségur »- c'est une expression que l'on entend souvent -, nous avons choisi en responsabilité, je le crois, de répondre aux problématiques spécifiques des professions concernées par une perte d'attractivité, chaque profession n'étant pas confrontée aux mêmes difficultés. C'est sur le fondement avéré de la perte d'attractivité des métiers que nous avons méthodiquement étendu les revalorisations à plusieurs reprises, au-delà de l'ambition initiale du Ségur. Vous le savez, deux protocoles d'extension avec les organisations syndicales ont été signés à l'issue d'une mission que le Premier ministre avait confiée à Michel Laforcade à propos des structures sanitaires, médico-sociales financées par l'assurance

Ce secteur est particulièrement marqué par des dérives lucratives : sous-effectif constant, dépenses réduites et, en conséquence, souffrance au travail du personnel soignant et accompagnant, qui se répercute sur les personnes âgées comme sur les familles.

en particulier dans ces établissements privés lucratifs ? Et dans quel délai ?

une inspection inopinée en 2018 à la suite de réclamations et de signalements qui avaient déjà été adressés à l'époque. Les révélations récentes laissent cependant penser que la situation était bien pire que ce dont nous avions alors connaissance.

sur lesquelles nous demandons au groupe Orpéa, dont le directeur général a été convoqué par Brigitte Bourguignon, de s'expliquer, là aussi, dans les plus brefs délais. Au-delà de cette situation particulière, je rappelle que le l'ensemble des soignants et des professionnels des établissements accueillant des personnes âgées. Dès 2018, nous avons installé une commission nationale pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance, qui rassemblait de nombreux experts. Elle a remis ses travaux au Gouvernement l'année dernière,

Nous connaissons la détresse des personnels, confrontés à des dilemmes éthiques inhumains : rester dans un secteur en manque de moyens constants pour prodiguer des soins décents ; ou bien le quitter alors même qu'il y a un manque de professionnels dans ces métiers. C'est le business : tout est rationalisé, jusqu'au rationnement des couches et des biscottes ! Des maisons de retraite sont rachetées par des multinationales et des fonds d'investissement, le tout avec de l'argent public ! Vous n'en avez pas dit un seul mot. L'une des grandes promesses d'Emmanuel Macron était de faire une loi structurante sur le grand âge ; celle-ci n'a jamais vu le jour. jour. Il nous faut un véritable service public du grand âge. Les Ehpad dépendant des groupes privés qui se sont rués vers l'or gris aux dépens de la qualité de vie de leurs patients doivent être mis sous tutelle. L'État ne doit plus laisser faire, car les personnes âgées ne sont pas des marchandises. Le grand âge doit sortir du marché La parole est à Mme Laurence Garnier, pour le groupe Les Républicains. groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur. Monsieur le ministre, Nantes a connu le week-end dernier un nouveau déferlement de violence urbaine. Vous avez annoncé hier l'engagement d'une procédure de dissolution du groupuscule d'ultragauche « Nantes révoltée » ; nous vous l'avions demandé avec la présidente de région et la députée de Nantes. C'est une bonne nouvelle. Je vous en remercie.

Les violences ont commencé avec le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Depuis, Nantes est devenue la capitale des manifestations ultraviolentes. Vous avez cédé aux zadistes en renonçant à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, donnant raison aux ultraviolents et envoyant le message politique irresponsable que la violence paye dans notre pays Je rappelle également que 95 % des manifestations à Nantes ne sont pas déclarées. Cela aussi, nous le dénonçons depuis des années. Ajoutez à cela la complaisance d'élus locaux encourageant l'ultragauche, qui défile aux cris de « Mort aux flics », et vous avez à Nantes le résultat que chacun connaît. Monsieur le ministre, pourquoi avez-vous attendu d'être à deux mois de l'élection présidentielle pour dissoudre un groupuscule qui détruit Nantes depuis des années ?

Monsieur le ministre, la réalité, vous la connaissez. Vous avez laissé Nantes s'enfoncer dans la violence. Les Nantais ne sont pas dupes de telles manoeuvres. Ils savent pertinemment que vous ne rattraperez pas en deux mois ce que vous n'avez pas fait pendant cinq ans. La

jamais les tensions entre la communauté enseignante et leur ministre n'ont été aussi fortes. Cette défiance est la pire ennemie de l'efficacité des politiques publiques. On vous a entendue sur la prétendue « dérive islamo-gauchiste » des universités. Mais, bizarrement, on ne vous a pas entendue sur le manque de moyens de ces Le Président de la République, lui, aurait trouvé une solution merveilleuse : faire payer les étudiants. Il me paraît insensé de penser que l'on va augmenter les moyens et le niveau des universités en faisant payer les étudiants ! Outre les moyens, le problème est en réalité celui de l'orientation l'inégalité d'accès à l'information sur les filières conduit à des taux d'échec record, notamment lors de la première année de licence. Comment est-il possible de faire peser la réussite des élèves uniquement sur le financement de l'université sans rompre le principe d'égalité ? C'est une erreur de penser que la gratuité est le problème. Le principal problème, c'est l'orientation, un problème intimement lié au manque d'information ; votre plateforme Parcoursup en est la preuve. C'est aussi pour cela que l'on retrouve toujours plus d'étudiants en première année de licence. Madame la ministre, ma question est simple : que comptez-vous faire pour l'orientation, afin que l'université soit un vrai choix

de passage de la première à la deuxième année de licence. Je vous le confirme, en 2017, nous avions atteint le record d'échecs. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer- je suis sûre que vous l'aviez remarqué -que nous avons augmenté de dix points

je pense que ce n'est déjà pas mal. Je puis vous l'assurer, sur le terrain, les gens commencent à voir la différence. Vous continuez à prétendre, alors que

pour nos concitoyens les plus démunis. Mis en place en loi de finances pour 2022 afin de geler l'augmentation des tarifs gaziers jusqu'au 1 juillet, ce dispositif offre une couverture louable face à l'augmentation de la demande mondiale et la restriction de l'offre. Il ne s'applique toutefois qu'aux habitations individuelles ou collectives justifiant d'une consommation inférieure à 150 mégawattheures et dotées d'un contrat réglementé gaz B1. Or ce sont des critères auxquels ne répondent malheureusement pas les bailleurs sociaux, chargés d'acheter le gaz en amont avant de le redistribuer à leurs locataires. Les organismes HLM vont ainsi subir de plein fouet la hausse des tarifs et n'auront d'autre choix que de répercuter celle-ci sur les factures de leurs locataires. Je parle ici non pas d'augmentations de quelques euros à la marge, mais bel et bien de hausses pouvant s'échelonner de 40 euros à 250 euros de provisions de charges supplémentaires par mois, et ce jusqu'à la fin de la saison de chauffe. C'est une ironie des plus mordantes lorsque l'on fait état des engagements pris par votre gouvernement pour protéger le pouvoir d'achat des Français ! Monsieur le Premier ministre, dans quels délais comptez-vous revenir sur ce dispositif, qui, s'il n'est pas rectifié de façon rétroactive, risque de mettre une fois de plus à l'amende nos concitoyens les plus fragiles ? La parole

qui vont ainsi voir leur pouvoir d'achat soutenu. Nous avons effectivement décidé- c'est une mesure nationale très forte -de geler les tarifs réglementés de l'électricité, en plafonnant leur hausse à 4 %, et les tarifs du gaz. La question que vous posez concerne les ménages qui n'achètent pas directement le gaz à un fournisseur à tarif réglementé, mais qui sont dans des contrats collectifs, en particulier ceux qui sont souscrits par les organismes de logements sociaux. Ces organismes de logements sociaux nous ont effectivement fait part voilà quelques jours à peine de difficultés, sachant qu'ils ne sont pas tous dans la même situation. Certains sont chauffés à l'électricité ou au réseau de chaleur. D'autres sont avec des contrats individuels pour les locataires, qui sont donc bien protégés. encore achètent eux-mêmes en contrat collectif le gaz, et ces contrats collectifs sont dans un certain nombre de cas eux-mêmes protégés, parce qu'indexés sur les tarifs réglementés, et dans d'autres cas, non.

pour peu que l'on passe en revue les cinq années de négligence à l'égard du logement social. Je pense aux coupes budgétaires opérées trois années de suite, au doublement de la TVA sur la construction de logements sociaux, à la très controversée réduction des APL au ralentissement sans précédent du rythme des constructions et, dernièrement, à la désindexation du plafond de ressources pour bénéficier de la réduction du loyer de solidarité. Nous savions qu'à vos yeux les maisons individuelles étaient devenues un « non-sens écologique ». Désormais, c'est l'habitat collectif à loyer modéré qui en prend pour son grade. Décidément, il ne sera pas exagéré de dire

avec son arme de service. Pierre avait 22 ans. Il était champion d'arts martiaux. Il était très apprécié par tous ses collègues et avait toute la vie devant lui. Avant ce geste désespéré, huit autres fonctionnaires de police ont mis fin à leurs jours depuis le 1 janvier : une hécatombe Je tiens à adresser au nom du groupe Union Centriste mes plus sincères condoléances à la famille de Pierre, à ses proches et à ses collègues, mais également à avoir une pensée pour tous les fonctionnaires de police, de gendarmerie, des douanes et de l'administration pénitentiaire qui ont mis fin à leurs jours ces dernières années. À chaque nouveau drame, il y a un nouveau message du Gouvernement et une émotion sincère. Mais après ? Qu'est-ce qui peut pousser un ou une fonctionnaire de police à commettre l'irréparable ? Telle est la vraie question qui doit être posée. Le manque d'effectifs, le vieillissement des matériels ou des locaux peuvent être des éléments qui constituent ce mal-être. Il est vrai que votre ministère a augmenté les effectifs et les moyens matériels alloués à la police et à la gendarmerie ; j'en ai eu la preuve dans mon département. Pourtant, ce mal-être et cette détresse sont toujours là ! Monsieur le ministre, on en arrive peut-être à ce geste ultime lorsque l'on considère que son travail perd petit à petit de son sens malgré la foi profonde que l'on a de la justice et de la défense de ses concitoyens.

Il était plein de jeunesse. Son geste touche bien entendu toute la police nationale, ses collègues de Marseille et pose des questions à l'administration qui le dirigeait. Si l'essentiel de ces suicides- et je ne dis évidemment

En 2019, mon prédécesseur avait mobilisé des moyens très importants pour pouvoir lutter contre les suicides dans la police nationale. J'ai décidé de les faire évaluer par une société de conseil extérieure.

de Paris a recommandé la fin du recrutement sur dossier pour les lycées Henri-IV et Louis-le-Grand, au profit d'une plateforme informatisée que tout le monde connaît, Affelnet.

Monsieur le sénateur, ce n'est pas la fin de la méritocratie scolaire Si ! C'est, au contraire, son rétablissement dans les lycées d'excellence. Nos objectifs sont clairs : en pleine cohérence avec l'esprit de l'école républicaine, nous l'équité, le mérite et rendre ces lycées potentiellement accessibles à tous les élèves parisiens, sur la base de leurs seuls résultats scolaires. C'est Madame la secrétaire d'État, votre argumentation pourrait se résumer en quelques mots : cachez ces bons élèves que je ne saurais voir ... Très bien ! Je comprends évidemment votre intention d'ouverture sociale, mais je réfute la corrélation entre le statut de boursier et les performances académiques d'un collégien. Je déplore l'abandon des parcours d'excellence dans l'enseignement public, ... Eh oui ! ... le constat de la « honte » de nos élites et

Sans être statisticiens, les Français constatent chaque jour, impuissants, la hausse des prix de nombreux produits de première nécessité. Pain, café, pâtes, sucre, fruits et légumes : les prix explosent, en particulier ceux de l'énergie et du carburant, qui a augmenté de 25 % en un an. Cette flambée des prix affecte particulièrement les Français aux revenus modestes, les plus fragiles, nos territoires ruraux et tous nos concitoyens qui sont contraints d'utiliser leur véhicule pour se déplacer et aller travailler. Pour répondre à la situation, le Premier ministre vient d'annoncer le relèvement de 10 % du barème de l'indemnité kilométrique. Un pansement sur une jambe de bois ! Cette proposition favorisera probablement moins de 5 % des foyers français, certainement parmi les plus aisés. les plus aisés. Les salaires stagnent, les retraites sont péniblement revalorisées de 1,1 %, les prix flambent. Le pouvoir d'achat des Français est en berne. Madame la ministre, que répondez-vous à tous ceux et toutes celles qui doivent, chaque jour, choisir entre manger, se chauffer ou faire le plein pour aller travailler ?

madame la ministre, mais je veux des réponses concrètes. Depuis des semaines, nous, socialistes, proposons une baisse de la TVA à 5,5 % sur les carburants pour soulager les Français, quitte à le faire de façon temporaire. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle ! L'urgence aujourd'hui est d'accompagner la sortie de crise des ménages, de tous ceux qui sont pris à la gorge par les hausses de prix. L'urgence, c'est aussi d'augmenter significativement les bas salaires, en particulier le SMIC. On ne peut avoir, d'un côté, le « quoi qu'il en coûte », et,

les organisations syndicales indiquaient qu'elles n'y étaient pas favorables et les organisations patronales faisaient part de leurs réserves. Toutes affirmaient néanmoins être d'accord pour renforcer le télétravail. Mme la ministre Élisabeth Borne confirmait elle-même qu'il existait un consensus sur le télétravail et qu'elle pouvait compter sur la responsabilité des employeurs et des salariés pour le renforcer. Néanmoins, le 28 décembre, coup de tonnerre ! Vous écrasiez la concertation et vous annonciez aux partenaires sociaux vouloir mettre en place des sanctions administratives pour les entrepreneurs qui ne respecteraient pas l'obligation du télétravail. Dans la foulée, toutes les organisations patronales jugeaient que ces amendes étaient une ineptie, alors que les entreprises avaient eu une conduite exemplaire depuis le début de la pandémie. Dans la foulée, nous vous indiquions combien cette idée était clivante et inopérante. Loin de nous écouter, vous avez continué à jeter l'opprobre sur une catégorie de Français, les chefs d'entreprise ... Surtout, alors que l'encre du projet de loi était à peine

à préciser avant la fin de l'année par un décret du Gouvernement la manière dont les sapeurs-pompiers pourront mettre en oeuvre les douze gestes techniques de secourisme et de soins ». En effet, la loi Matras offre à nos sapeurs-pompiers la possibilité de dispenser des actes de soin d'urgence,

qu'attendez-vous ? Par ailleurs, les quatre rapporteurs du texte à l'Assemblée nationale et au Sénat, dont je fais partie, ont pris la peine de vous écrire afin de vous éclairer sur le sens que le législateur entend donner à ces dispositions. Sachez, monsieur le Premier ministre, que, si le décret à venir ne respectait pas la lettre de la loi, nous inviterions les présidents de SDIS à saisir le Conseil d'État afin que le décret soit annulé. Et si celui-ci respectait la lettre de la loi, mais en dénaturait l'esprit, nous modifierions la loi afin de le rendre caduc. Très bien ! Enfin, je souhaiterais obtenir des explications sur l'absence de revalorisation des indemnités que perçoivent les SDIS lorsqu'ils assurent des carences ambulancières à la demande des SAMU. Là encore, malgré les promesses présidentielles, toujours rien ! Il n'y a pourtant : il s'agit de modifier un chiffre dans un arrêté ... Mais peut-être attendez-vous l'étude d'un cabinet de conseil pour procéder à cette modification ... On n'est jamais trop prudent Monsieur le Premier ministre, les pompiers méritent vraiment mieux que des paroles en l'air, mieux que de la communication stérile, mieux que des discours de Sainte-Barbe. Il est grand temps d'agir

Françoise Dumont, pour la réplique. Vous aviez imposé un calendrier contraint au Parlement pour que le Président de la République puisse faire des annonces au congrès des sapeurs-pompiers. Encore une fois, vous êtes dans la communication, et non dans l'action

La séance est reprise. Mes chers collègues, sur la proposition du groupe de travail sur la modernisation des méthodes de travail du Sénat, la conférence des présidents a décidé qu'un débat d'actualité se tiendrait lors de chaque semaine de contrôle, après la séance de questions d'actualité au Gouvernement. La conférence des présidents a inscrit le premier débat d'actualité mercredi 2 février. Après concertation avec les groupes politiques, ce débat pourrait porter sur le thème : « Énergie et pouvoir d'achat : quel impact de la politique du Gouvernement ? » et aurait lieu sous forme de discussion générale. Y a-t-il des observations ? Il en est ainsi décidé. Par ailleurs, par lettre en date de ce jour, M. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains, demande le retrait de l'ordre du jour du mardi 1 février de la proposition de loi tendant à expérimenter un chèque emploi petites communes pour l'emploi d'agents contractuels et vacataires. En conséquence, nous pourrions avancer le débat sur le thème : « Quelle politique ferroviaire pour assurer un maillage équilibré du territoire ? » à la suite du débat sur les menaces que les théories du wokisme font peser sur l'université, l'enseignement supérieur et les libertés académiques. Le début du débat sur le suivi des ordonnances serait quant à lui décalé à dix-huit heures. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé. Par lettre en date du 25 janvier, M. Hervé Marseille, président du groupe Union Centriste, demande le retrait de l'ordre du jour de l'espace réservé à son groupe du mercredi 2 février de la proposition de loi visant à améliorer la prise en charge des personnes atteintes du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il demande l'inscription à la place de ce texte d'un débat sur le thème : « L'amélioration de la prise en charge des personnes atteintes du trouble du déficit de l'attention. » Acte est donné de cette demande. Ce débat se tiendrait sous la forme d'une discussion générale d'une heure. Y a-t-il des observations ? Il en est ainsi décidé. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein des commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte et de la proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. L'ordre du jour appelle l'examen du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer relatif au siège de l'Agence de l'Union européenne

sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission mixte paritaire (CMP) est parvenue, le 5 janvier dernier, à un texte commun sur le projet de loi de ratification de l'ordonnance du 21 avril 2021 sur la représentation des travailleurs de plateformes. Ce texte a pour objet d'organiser un dialogue social entre les plateformes numériques et les travailleurs indépendants y ayant recours dans deux secteurs qui cristallisent le débat sur les questions de statut et de protection de ces travailleurs : la conduite de véhicule de transport avec chauffeur (VTC) et la livraison de marchandises en véhicule à deux ou trois roues. Tout en regrettant la méthode suivie par le Gouvernement, qui choisit de passer par une nouvelle ordonnance pour compléter le cadre de ce dialogue social, et en observant les évolutions concomitantes du contexte européen, le Sénat avait globalement approuvé l'objectif de faire émerger des garanties collectives en faveur des travailleurs des plateformes par la voie de la négociation. Un accord répondant aux préoccupations du Sénat a ainsi pu être trouvé sur ce texte à l'issue d'échanges constructifs avec la rapporteure de l'Assemblée nationale, Carole Grandjean, que je remercie sincèrement de l'écoute Le Sénat avait approuvé la ratification de l'ordonnance du 21 avril 2021 sous réserve de quelques modifications. Deux amendements du Sénat relatifs à la nouvelle Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, l'ARPE, ainsi repris dans le texte de la CMP. D'une part, l'objet de cet établissement public restera circonscrit à la régulation du dialogue social- et non pas des relations sociales -entre les travailleurs et les plateformes des deux secteurs concernés. D'autre part, est confirmée la suppression de la présence d'un député et d'un sénateur au conseil d'administration de cet établissement public sous tutelle de l'État, en cohérence avec la volonté du Sénat de rationaliser les organismes extraparlementaires, même si ce point a fait débat jusqu'à hier soir. En revanche, il a semblé préférable de renoncer au droit d'option que le Sénat avait prévu concernant les travailleurs qui seraient électeurs dans les deux secteurs d'activité, car sa mise en oeuvre se serait écartée du droit commun applicable aux salariés et aurait pu engendrer des freins opérationnels à l'organisation des premières élections. le Sénat s'était efforcé d'opérer un tri afin de restreindre l'habilitation à prendre une nouvelle ordonnance aux dispositions apparaissant comme les plus urgentes ou techniques. Il avait notamment supprimé tous les éléments de l'habilitation concernant l'organisation d'un dialogue social au niveau de chaque plateforme, considérant que les principaux enjeux en matière de régulation de l'économie des plateformes se situaient au niveau sectoriel et que la mise en place d'un dialogue social de plateforme interviendrait éventuellement dans un second temps. Ces modifications ont été maintenues dans le texte de la CMP, ce qui représente, de mon point de vue, une garantie importante. Le Sénat avait, en conséquence, fixé la durée de l'habilitation à six mois, le délai de douze mois prévu par l'Assemblée nationale nous ayant paru excessif pour la mise en place du seul dialogue social de secteur. Sur ce point, la CMP a adopté une position intermédiaire, en fixant à neuf mois le délai pour prendre les ordonnances. Le Sénat avait par ailleurs supprimé les alinéas visant à confier à l'ARPE, d'une part, un rôle de médiation entre plateformes et travailleurs, et, d'autre part, un rôle d'expertise, d'analyse et de proposition concernant l'activité des plateformes et de leurs travailleurs. Le texte de la CMP réintègre ces alinéas en tenant compte des réserves du Sénat : le rôle de médiation de l'ARPE ne concernera ainsi que les relations entre les représentants des travailleurs et les plateformes, et son rôle d'expertise s'exercera dans le cadre de sa mission de régulation du dialogue social. Enfin, le Sénat avait souhaité inscrire directement dans le projet de loi les règles concernant les thèmes et la périodicité de la négociation obligatoire sectorielle. Il avait ainsi précisé à l'article 3, en lieu et place de l'habilitation de l'article 2, que les organisations représentatives au niveau d'un secteur devraient obligatoirement négocier, selon une périodicité fixée par accord collectif et au moins tous les quatre ans, sur trois thèmes structurants communs aux deux secteurs : la fixation du prix des prestations, le développement des compétences professionnelles et la prévention des risques professionnels. Il n'a pas été possible d'aboutir à une rédaction commune de ces dispositions, en raison notamment des incertitudes qui demeurent sur leur compatibilité avec le droit européen de la concurrence. La CMP les a donc rétablies à l'article 2 sous la forme d'une habilitation, dont le champ a été précisé : il est clairement inscrit que les thèmes de négociation doivent notamment inclure les trois thèmes identifiés par le Sénat. L'article 3 a, en cohérence, été supprimé. Au total, malgré sa forme contestable et les incertitudes qui demeurent, notamment du fait du lancement d'un chantier législatif au niveau européen, le texte ouvre une voie de régulation prometteuse pour les secteurs concernés afin d'améliorer les protections, aujourd'hui insuffisantes, dont bénéficient les travailleurs indépendants, et ce sans compromettre les bénéfices économiques offerts par le développement des plateformes. Mes chers collègues, je vous invite donc aujourd'hui, au nom de la commission mixte paritaire, à adopter ce projet de loi. Très bien

d'État. Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame le rapporteur Frédérique Puissat, mesdames, messieurs les sénateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi « Travailleurs des plateformes ». Le 5 janvier dernier, cette commission aboutissait à un accord sur ce texte, après une première lecture à l'Assemblée nationale, en septembre, et au Sénat, en novembre. Je tiens à remercier particulièrement les membres de la CMP des deux assemblées. Ce travail collectif a permis d'aboutir à un texte ambitieux et équilibré, qui, conformément à l'engagement du Gouvernement, fournit un socle de droits nouveaux aux travailleurs des plateformes. C'était, en quelque sorte, votre conclusion, madame le rapporteur. Ce texte repose sur une conviction : la négociation collective est la meilleure méthode pour bâtir une protection sociale adaptée aux travailleurs des plateformes. Je rappelle que le premier objectif de ce projet de loi est de ratifier l'ordonnance du 21 avril dernier, consistant à faire émerger un dialogue social dans le secteur des plateformes de mobilité. Cette ratification est une première pierre posée en vue de la construction d'une véritable démocratie sociale dans le secteur, ce dont nous pouvons nous réjouir collectivement. Avec elle, nous voulons accompagner le développement des plateformes de mise en relation, tout en veillant à mieux protéger leurs travailleurs. proposer les conditions d'un dialogue social structuré entre les plateformes et les travailleurs qui y recourent, afin de construire des droits nouveaux- rémunération minimale, formation professionnelle, santé au travail, un sujet qui m'est cher tout en respectant l'indépendance à laquelle nombre d'entre eux sont attachés. Il s'agit aussi d'adapter le droit du travail aux nouvelles formes d'emploi. s'inscrit dans la continuité d'un travail de réflexion et de concertation approfondi, mené d'abord par Jean-Yves Frouin, puis par Bruno Mettling, que je tiens tous deux L'ordonnance du 21 avril dernier prévoit l'organisation d'une élection nationale, permettant aux près de 100 000 travailleurs des deux secteurs d'activité concernés, c'est-à-dire les chauffeurs de VTC et les livreurs à vélo, d'élire leurs représentants. Cette élection, qui se tiendra du 9 au 16 mai 2022, leur permettra d'accéder pour la toute première fois à une représentation syndicale. Sa réussite est au coeur des missions confiées à la nouvelle instance de facilitation du dialogue social, également prévue par cette ordonnance

Cette installation, mesdames, messieurs les sénateurs, est une première étape importante. Elle marque notre volonté de voir se déployer rapidement les dispositions du projet de loi que vous êtes appelés à voter aujourd'hui. Au-delà de l'organisation des élections, cette jeune autorité sera chargée d'accompagner les nouveaux représentants pour la réussite des premières négociations qui seront lancées. En effet, l'ARPE a vocation à devenir un facilitateur du dialogue social, en même temps qu'un observatoire des évolutions de l'activité du secteur des plateformes. ce stade, je veux saluer les avancées importantes permises sur ce texte par les deux chambres parlementaires, qui ont complété utilement les missions attribuées à cette autorité. Mme le rapporteur l'a rappelé à l'instant, mais j'y reviens succinctement. Dans ce projet de loi, deux nouveaux rôles lui ont ainsi été confiés : un rôle de reconnaissance des organisations représentatives des plateformes et un rôle de médiation en cas de différends entre les plateformes et les représentants des travailleurs. L'enrichissement de ses missions permettra à l'ARPE d'accroître rapidement sa crédibilité et de gagner en efficacité. Par ailleurs, le travail de la commission mixte paritaire a permis de préciser et de mieux définir les rôles d'expertise et de médiation dévolus à ce nouvel établissement public administratif, de sorte qu'il pourra prendre rapidement la mesure de son portefeuille et monter pleinement en puissance. Au-delà de ces avancées, ce texte ouvre la voie à de nouveaux travaux législatifs, qui permettront de finaliser les modalités du futur dialogue social dans ce secteur. C'est tout le sens de l'article 2, qui vous demande d'habiliter le Gouvernement à approfondir, par voie d'ordonnance, le cadre de la négociation collective entre les représentants des plateformes et de leurs travailleurs. Le recours à cette procédure répond à un impératif d'efficacité, qui rend nécessaire de finaliser le cadre de ce dialogue social avant la tenue des élections professionnelles au mois de mai, pour donner de la visibilité aux travailleurs des plateformes. Je veux, à ce sujet, saluer le compromis obtenu quant à la définition des thèmes qui seront ouverts à la négociation collective. En faisant le choix de renvoyer cette liste de thèmes à la future ordonnance, l'Assemblée nationale et le Sénat démontrent, une fois encore, que leur travail de coconstruction est essentiel pour aboutir à des dispositifs équilibrés et utiles. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l'aurez compris, ce texte de compromis pose les jalons d'un dialogue social dans le secteur des plateformes de mobilité. Nous pouvons en être fiers. Nous sommes convaincus que cette méthode permettra de bâtir des protections nouvelles, répondant du mieux possible aux aspirations de près de 100 000 travailleurs indépendants.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, notre droit doit s'adapter en permanence aux évolutions d'un monde économique qui se transforme. Ainsi, le sujet de la protection des travailleurs liés à des plateformes numériques est devenu la préoccupation du législateur, conduisant notre Haute Assemblée à approfondir sa réflexion par la rédaction de plusieurs rapports. si la mise en relation de travailleurs, de plateformes et de consommateurs crée de nouveaux services et des opportunités d'emplois, elle vient bouleverser les règles sociales habituellement attachées à l'exercice d'une profession salariée ou indépendante. Cela est particulièrement vrai dans les deux secteurs de la conduite de VTC et de la livraison de marchandises en véhicule à deux ou trois roues, les travailleurs en relation avec des plateformes y étant exposés à des risques particuliers et à une certaine précarité. De plus, l'asymétrie des pouvoirs dans l'organisation des activités impose une vigilance particulière. Le présent texte est particulièrement important, car il privilégie la voie du dialogue social pour assurer la protection des travailleurs des deux secteurs, au-delà de la question de leur statut juridique, qui semble, elle, devoir évoluer au niveau européen, comme l'a souligné notre rapporteur. Je me réjouis que nous soyons parvenus à un accord avec les députés, lors d'une commission mixte paritaire conclusive à laquelle j'ai participé. le cadre de leur rapport sénatorial, nos collègues Frédérique Puissat, Catherine Fournier et Michel Forissier recommandaient, comme je l'avais souligné en première lecture, le développement de ce dialogue social au travers d'une meilleure représentation des travailleurs et des plateformes. Ils prévoyaient par ailleurs des thèmes de négociation obligatoires, tels que la détermination des revenus des travailleurs, le développement de leurs compétences, la prévention des risques professionnels,

C'est à cette condition que le Sénat a pu accepter l'habilitation donnée au Gouvernement pour fixer par ordonnance la définition des thèmes débattus et la périodicité de la négociation. J'en profite pour saluer le travail de notre rapporteur, dont les connaissances et le sens de l'écoute ont été fort utiles pour améliorer ce texte. En vertu de la rédaction proposée par le Sénat, l'habilitation porte sur l'organisation du dialogue social au niveau de chaque secteur, et non au niveau de chaque plateforme, ce qui aurait été prématuré et pourra être mis en place ultérieurement. ultérieurement. Notre Haute Assemblée a également mieux encadré les missions de l'ARPE, autorité créée pour organiser les élections professionnelles et accompagner le dialogue social. Nous avons souhaité recentrer son rôle sur la régulation de ce dialogue entre travailleurs et plateformes plutôt plutôt que sur la régulation de leurs relations sociales. La CMP a également suivi nos propositions en encadrant les pouvoirs de médiation de l'ARPE, ainsi que ses activités d'expertise. Enfin, comme nous souhaitions éviter toute perte de temps dans l'organisation du dialogue social de ce secteur, nous avons retenu un délai de neuf mois pour la durée d'habilitation, délai plus avantageux que les douze mois initialement prévus par les députés, mais moins exigeant que les six mois que nous avions prévus en première lecture. Rappelons que le Gouvernement disposait de dix-huit mois dans le texte initial. Ainsi le présent texte a-t-il été particulièrement enrichi par nos travaux. L'étape fondamentale franchie aujourd'hui repose sur le poids donné à la négociation collective. Nous souhaitons que cette voie de régulation soit féconde, et qu'elle puisse par la suite être une source d'inspiration pour d'autres pays. Aussi notre groupe votera-t-il ce projet de loi. La parole

depuis la loi El Khomri, qui accordait aux travailleurs des plateformes le droit de créer une organisation syndicale, une loi était nécessaire pour l'organisation du dialogue social en leur sein. Était attendu,, un un cadre légal permettant un progrès significatif dans les conditions de travail souvent indignes de ces travailleurs, un cadre s'appuyant notamment sur le droit commun et les dispositions du code du travail.

Après la promulgation de ce texte, les travailleurs des plateformes n'auront toujours pas de salaire minimum garanti, toujours pas de protection contre les licenciements par déconnexion de la plateforme, toujours pas d'encadrement de la durée maximale de travail, toujours pas de congés ni de jours de repos sanctuarisés et rémunérés. Le texte sur lequel le Sénat et l'Assemblée nationale se sont accordés propose une légère compensation de ces manques à l'article 2, lequel dispose que le dialogue social mené avec les plateformes devra comprendre la fixation du prix des prestations, le développement des compétences professionnelles et la prévention des risques professionnels. en renvoyant ces droits sociaux à la négociation collective, nous autorisons la création d'un droit du travail différencié, qui a toutes les chances de se montrer moins disant, car rien n'est fait par ailleurs pour corriger les inégalités nées du rapport de force entre les plateformes et les travailleurs. Le dialogue social ne peut améliorer la situation des travailleurs d'une branche, quelle qu'elle soit, que si la puissance publique impose une base de négociation protectrice, en l'occurrence celle proposée par le code du travail, dont une des fonctions est de rééquilibrer le rapport de subordination entre l'employeur et les travailleurs. lien de subordination a été reconnu par plus d'une centaine de décisions de justice en Europe. Après une résolution du Parlement européen allant dans ce sens, la Commission européenne a présenté en décembre dernier une directive sur la présomption de salariat pour tous les travailleurs des plateformes. La Commission considère précisément que c'est le statut erroné d'indépendant qui empêche ces travailleurs de jouir des droits sociaux auxquels ils devraient sans cela avoir droit : salaire minimum, réglementation du temps de travail, protection sociale. C'est donc le statut et le renvoi aux droits sociaux qui lui sont attachés qui protège les travailleurs, et non une prétendue autorégulation du dialogue social de parties placées dans des situations inégales, bien souvent synonyme de régression sociale. Dans la documentation qui accompagnait son introduction en Bourse en 2019, Uber écrivait, page 30 : « Étant donné que nous prévoyons de réduire les incitations monétaires des conducteurs afin d'améliorer nos performances financières, nous nous attendons à ce que leur insatisfaction augmente ».

De fait, si Uber insiste tant sur l'indépendance de ses chauffeurs, c'est que leur requalification en salariés représenterait un surcoût significatif de l'ordre de 20 % à 30 %. La préservation des profits de cette firme tient donc entièrement sur la promesse mensongère de l'autonomie des travailleurs, renforcée par ce texte. En effet, à l'Assemblée nationale, la rapporteure a précisé dans son rapport que l'objectif des dispositions, maintenues aux alinéas 16 et suivants de l'article 2 du texte de la CMP, était de « réduire le faisceau d'indices susceptibles de révéler l'existence d'un lien de subordination, tel que celui-ci est défini par la jurisprudence de telle sorte que " les risques de requalification de leur contrat commercial en contrat de travail " soient limités ». Le but est donc de sécuriser les plateformes

200 000 travailleurs en dehors de tout cadre légal, qui leur permettrait de se défendre équitablement face au management algorithmique, et nous privons la sécurité sociale d'importantes ressources. Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ne votera pas ce texte. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

voici donc un dialogue social vidé de sa substance. Pour un autre avenir en faveur des travailleurs des plateformes numériques, plusieurs groupes politiques, dont le CRCE, ont, en plusieurs occasions, proposé des mesures concrètes, jamais votées par le Sénat. Qu'avons-nous eu en retour de la part du Gouvernement depuis cinq ans ? Des textes d'une inefficacité navrante, et ce projet de loi n'y change rien. Bien plus grave, il vient consacrer la valeur travail comme une valeur malléable en fonction des modèles économiques, quelle que soit leur rentabilité. Elle serait aménageable selon la qualité des travailleurs, qualifiés ou non, ou selon la qualité estimée des prestations effectuées. On aurait un statut d'indépendant qui serait différent selon que vous êtes travailleur économiquement dépendant de plateforme ou que vous êtes travailleur indépendant choisi. Le premier se verrait privé d'autonomie et serait corvéable à merci quand le second pourrait négocier librement ses prix et les caractéristiques de sa prestation. Quelle contradiction ! Mes chers collègues de la partie droite de l'hémicycle ont voté à l'unanimité le rapport d'information sur l'« ubérisation » de la société, alertés par le risque de « plateformisation » de la société par les secteurs traditionnels ou les fonctions libérales. Seulement, au moment de réguler les plateformes numériques de travail, ils se sont retrouvés embarrassés devant l'avantage et le confort qu'il y a à trouver une petite main plus vite et pour moins cher. Pour que le rouage de la servitude continue de tourner, il faut donc que le Gouvernement préserve le contrôle des plateformes de travail sur leurs travailleurs, tout en se dégageant d'une quelconque responsabilité. Lors de l'adoption de ce texte en première lecture dans cet hémicycle, nous avions, à l'article 3, contraint chaque secteur à négocier certains thèmes, dont la fixation des prix. Pourquoi cela a-t-il disparu de la version finale ? ! Le Président de la République a pourtant annoncé au Parlement européen que la création d'un SMIC européen était une priorité. Pourquoi alors refuser qu'une rémunération minimale soit l'objet du dialogue ? Si des indépendants peuvent normalement négocier leurs prix, on consacre ici le fait que tel n'est pas le cas pour ceux des plateformes. On officialise ainsi l'indépendance contrainte et l'autonomie à deux vitesses. 4 de l'article 2, il y a, parmi les thèmes de négociation obligatoire, « les modalités de détermination des revenus des travailleurs ». Comprenez la subtile manoeuvre : c'est une chose d'imposer de se mettre d'accord sur une rémunération minimale, c'en est une autre d'imposer de discuter de la manière dont les revenus sont calculés par la plateforme. Même contradiction à l'alinéa 18 de l'article 2 : « en leur garantissant une marge d'autonomie pour déterminer les modalités de réalisation des prestations » ... mais pas des prix ! Autonome, mais, quand même

autorise la rupture du contrat commercial des représentants désignés en application de l'article L. 7343-13 ». Une autorité administrative qui se prononce sur un contrat commercial ... Vous êtes sûrs ? On voit bien que cela a été pensé en dehors de toute objectivité. C'est pratique, quand on est déjà poursuivi pour travail dissimulé ... Et que dire des conditions de représentativité, d'une complexité kafkaïenne, qui feront gagner du temps aux plateformes plus qu'elles n'entraîneront l'adhésion des travailleurs ? Enfin, il est légitime d'interroger l'opportunité de ce texte au regard de la proposition de la Commission européenne, qui, elle, porte une ambition en instaurant une présomption réfragable de relation de travail, allant ainsi dans le sens des décisions de justice européennes.

sur un texte visant à organiser un dialogue social entre les plateformes numériques et les travailleurs indépendants qui y ont recours. Ces dernières années ont vu l'émergence des plateformes numériques de mise en relation, qui ont offert une activité professionnelle à de nombreux travailleurs, principalement des jeunes sans formation et éloignés de l'emploi. Si nous pouvons nous réjouir que ce public accède ainsi à un travail, il n'en reste pas moins qu'il convient de regarder avec attention les conditions dans lesquelles ces activités professionnelles sont réalisées. Je note que le législateur, à la faveur de plusieurs travaux d'expertise, à la suite d'initiatives parlementaires, n'a pas manqué de « flécher » certaines limites de ce type d'activités. Pour autant, notre corpus juridique n'est pas resté sans modification

Si le présent projet de loi ne présente aucune mesure législative concernant l'amélioration des conditions de travail, pas plus que sur la santé des salariés des plateformes, il permettra, avec la ratification de l'ordonnance d'avril 2021,

précisions cruciales, comme la redéfinition du périmètre de l'ARPE. Nous pouvons encore une fois nous réjouir de cette recherche de consensus. Aussi, je vous appelle, mes chers collègues, à soutenir un texte qui s'inscrit dans la lignée de la loi du 8 août 2016, a inscrit le principe de la responsabilité sociale des plateformes à l'égard des travailleurs indépendants. Avant d'en terminer, je me permettrai d'interpeller le Gouvernement, monsieur le secrétaire d'État. En consultant le Parlement sur l'ordonnance hasardeuse d'avril 2021, en vous proposant simplement d'instituer un dialogue social entre travailleurs indépendants et plateformes, vous avez, contre votre volonté, réveillé l'ardent besoin de recourir au code du travail, de rétablir la place de l'État face aux géants de l'ubérisation et de croire encore aux vieux principes du rapport de force. En vous frottant à l'univers du dialogue social, vous avez élevé la température de l'ancien monde, qui, d'ailleurs, n'a jamais été autant d'actualité. La Commission européenne proposait, en décembre dernier, la présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes. Les Pays-Bas, la Belgique, l'Angleterre et la Californie ont multiplié les arguments en faveur de la qualification de « salariat » pour ces travailleurs. Enfin, la Cour de cassation a contredit le Gouvernement dans deux arrêts. Le choix du Gouvernement de recourir aux ordonnances vous oblige et vous condamne à passer les étapes si vous ne voulez pas que ce texte reste à l'état de calmant destiné à bercer d'illusions des milliers de faux travailleurs indépendants dans la misère. Monsieur le secrétaire qu'en matière de régulation et de maîtrise du fait numérique les choses avancent. Le volet numérique du discours du Président de la République, la semaine dernière, devant le Parlement européen, ainsi que la taxation des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) laissent à penser, et à espérer, que nous en viendrons un jour à obliger les plateformes à rendre leurs algorithmes En présidant l'Europe, la France doit désormais se hisser à la hauteur de sa responsabilité historique en prenant ce sujet à bras-le-corps, bien qu'elle ait déjà du retard sur ses partenaires. En tout état de cause, le groupe Union Centriste votera favorablement ce texte. La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis a pour objet de réguler les relations sociales entre les plateformes numériques et les travailleurs indépendants. Il est vrai que l'émergence de ces plateformes et, avec elle, l'apparition d'une nouvelle organisation du travail, nous amènent à nous interroger, notamment, sur le statut de ces travailleurs ou sur leurs droits sociaux. En somme, nous devons désormais prendre en compte le modèle économique de ces plateformes, afin de mieux protéger et de garantir suffisamment les droits des travailleurs qui y ont recours. Le débat sur la détermination du cadre des rapports entre les plateformes numériques et les travailleurs ayant opté pour la microentreprise n'est pas nouveau. En effet, le législateur a déjà fait oeuvre de régulation à plusieurs reprises, afin de rétablir un équilibre dans les relations qui lient ces travailleurs indépendants aux plateformes numériques.

déterminant les droits et les obligations des plateformes, ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elles sont en relation. Dans la continuité de ces textes, et sans remettre en cause les statuts existants, le présent projet de loi a pour ambition de renforcer les droits des travailleurs indépendants, en permettant notamment de faire émerger des garanties collectives en faveur des travailleurs des plateformes par la voie du dialogue social. Avant de poursuivre, il convient de rappeler que le développement de ces plateformes numériques est généralement considéré comme l'opportunité d'exercer une activité professionnelle pour de jeunes travailleurs sans formation et n'ayant parfois aucune expérience du monde du travail. L'ubérisation croissante d'une partie de notre mode vie, qui s'est accélérée avec la crise sanitaire, nous amène à réfléchir à notre modèle social, car tout laisse à croire que ce modèle économique s'étendra probablement à d'autres secteurs d'activité. Il est donc nécessaire et urgent de fixer un cadre légal clair pour éviter toute précarisation du travail. Il est nécessaire de construire un dialogue social entre les plateformes et les travailleurs indépendants. Je partage le point de vue de M. le secrétaire d'État sur ce sujet. C'est pourquoi, dans son rapport de mai 2020 sur le droit social applicable aux « travailleurs indépendants économiquement dépendants », la commission des affaires sociales du Sénat avait déjà formulé des recommandations, afin de dépasser le débat sur le statut de ces travailleurs et de développer leurs droits de manière pragmatique, notamment par la voie du dialogue social. social. Dans ce contexte, la commission des affaires sociales est restée fidèle à ses propositions lors de la préparation de ce projet de loi. Je tiens aussi à féliciter tous nos collègues qui ont participé à la commission mixte paritaire de la qualité du travail effectué. que l'article 1 du projet de loi vise à ratifier, permet aux travailleurs indépendants des plateformes de mobilité de désigner leurs représentants pour 2022. Par ailleurs, on ne peut que saluer la création d'une Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE) ce nouvel établissement public aura pour rôle de réguler les relations entre les deux parties. Mes chers collègues, ces dispositions ne constituent qu'une première étape dans l'élaboration d'un cadre permettant le développement du dialogue social entre les travailleurs indépendants et les plateformes, lesquelles peuvent encore être améliorées, comme tout texte législatif.

d'un tiers-statut pour les travailleurs des plateformes, alors même que le risque d'expansion du phénomène d'ubérisation pèse sur un nombre croissant de secteurs d'activité. L'idée d'un tiers-statut recule dans la plupart des pays européens, à la suite de la multiplication des décisions de justice reconnaissant le lien de subordination des travailleurs de ces plateformes, comme cela a été le cas en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, en Allemagne ou encore, récemment, aux Pays-Bas. Jean-Yves Frouin a également clairement écarté ce statut dès décembre 2020, en proposant de salarier les travailleurs des plateformes le portage salarial ou une coopérative d'activité et d'emploi. C'est cette seconde option que nous préconisons depuis plusieurs années, afin de sécuriser la relation juridique des travailleurs tout en leur apportant de l'autonomie- ils y sont attachés -dans l'exercice de leur activité l'exercice de leur activité et en développant un modèle de plateforme numérique plus vertueux, s'inscrivant dans l'économie sociale et solidaire. La proposition de loi de notre groupe visant à lutter contre l'indépendance fictive, portée par Olivier Jacquin et dont je fus le rapporteur, prévoyait en outre des mesures adaptées et efficaces. Elle prévoyait, premièrement, la création d'une action de groupe au profit des travailleurs de plateformes, qui permettrait de les requalifier en tant que salariés ; deuxièmement, l'instauration d'une présomption de salariat dès lors que la majeure partie du revenu est issue de l'exploitation d'un algorithme, la charge de la preuve se trouvant ainsi inversée inversée ; troisièmement, la capacité pour les conseils de prud'hommes de se prononcer sur les demandes de requalification et d'exiger la production des algorithmes utilisés. Je rappelle que ces solutions sont déjà mises en oeuvre dans d'autres pays européens, notamment en Espagne, et qu'elles sont préconisées par le Parlement européen, ainsi que par la Commission européenne dans la proposition de directive qu'elle a présentée le 9 décembre dernier. vise à garantir la bonne détermination du statut professionnel des travailleurs de plateformes par le biais d'une présomption de salariat, pour laquelle elle fixe des critères d'appréciation. Elle inverse à son tour la charge de la preuve : il reviendra à la plateforme qui contesterait le statut de salarié de prouver qu'il n'existe pas de relation de salariat. La Commission européenne fait ainsi clairement le choix du salariat, conformément au positionnement du Parlement européen et aux revendications des syndicats, et rejette le tiers-statut. Elle propose en outre de renforcer la transparence dans l'utilisation des algorithmes par les plateformes de travail numériques et de créer le droit pour les travailleurs de contester des décisions automatisées.

et les plateformes à l'échelon sectoriel. Cet article intègre une partie des dispositions de l'article 3, qui a été supprimé, en prévoyant que l'ordonnance définira les thèmes et la périodicité de la négociation obligatoire. Parmi ces thèmes figurent les modalités de détermination des revenus des travailleurs. Le Conseil d'État estime à cet égard que ce sera d'application incertaine, l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne permettant pas à des indépendants de dialoguer entre eux concernant leur rémunération. La question de la constitutionnalité de cette disposition peut donc être posée. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre les conclusions de la commission mixte paritaire sur ce projet de loi et rappelle qu'il est urgent d'améliorer la protection de ces travailleurs précaires, qui sont malheureusement de plus en plus nombreux dans notre pays. La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 5 janvier dernier est donc parvenue à un accord sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance relative aux modalités

Ce texte était attendu. Il est en effet urgent, dans la lignée de la loi relative au travail et de la loi d'orientation des mobilités, de faire évoluer le cadre juridique qui gouverne les relations professionnelles entre les plateformes et les travailleurs indépendants, en particulier dans le secteur des voitures de transport avec chauffeur et dans celui de la livraison de marchandises. Le développement exponentiel de ces plateformes et l'augmentation du nombre de travailleurs qui y ont recours appelaient en effet une réponse rapide. Seul un dialogue social renforcé est à même d'assurer à 50 000 travailleurs les droits et la souplesse que leur statut d'indépendant leur garantit. L'ordonnance du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation qu'il nous est proposé de ratifier est une pierre de plus que nous apportons à l'édification d'un cadre protecteur pour ces nouveaux travailleurs. crée l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, un nouvel établissement public chargé de réguler les relations sociales entre plateformes et travailleurs indépendants. Elle prévoit également une élection nationale, à tour unique et par vote électronique, organisée afin de permettre aux travailleurs indépendants de désigner les organisations qui les représenteront. Ce scrutin aura lieu du 9 au 16 mai prochain. C'est un premier pas historique. À l'article 1, la commission mixte paritaire a jugé préférable de ne pas imposer aux travailleurs qui exercent une activité de conduite de VTC et de livraison de marchandises de choisir un secteur plutôt qu'un autre pour exercer leur droit de vote. de vote. Elle a estimé que cette solution présentait le risque de complexifier l'organisation des élections. L'accord recentre par ailleurs la mission de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

mission d'expertise, d'analyse et de proposition concernant l'activité des plateformes et des travailleurs. Conformément à la volonté du Sénat, qui jugeait ces dispositions prématurées, la commission a supprimé à l'article 2 les éléments de l'habilitation relatifs à l'organisation d'un dialogue social à l'échelon des plateformes pour ne conserver qu'un dialogue social de secteur. Le Sénat et l'Assemblée nationale, attachés à encadrer davantage les futures dispositions relatives au champ de la négociation collective l'échelle des secteurs, se sont par ailleurs entendus pour que l'habilitation définisse plus précisément les thèmes et la périodicité de cette négociation, sans qu'il soit nécessaire de conserver l'article 3.

afin que les premières élections des représentants des travailleurs des plateformes puissent avoir lieu dans les meilleures conditions. Considérant le travail accompli par nos deux chambres, mais également le fait que ce projet de loi de ratification et d'habilitation est une étape indispensable,

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en 2017, le verbe « ubériser » faisait son entrée dans nos dictionnaires, avec la définition suivante Déstabiliser et transformer, avec un modèle économique innovant tirant parti des nouvelles technologies ». Depuis bien des années désormais, nous pouvons observer les conséquences de l'ubérisation de notre société. Au départ, nous avons suivi la montée en puissance des VTC et le développement des premières applications. Depuis lors, les plateformes numériques se sont saisies de la livraison dans le domaine de la restauration. Elles connaissent un essor impressionnant depuis 2020 et le début de la pandémie que nous vivons toujours. Toutefois, les transports et la nourriture ne sont pas les seuls secteurs économiques atteints par ce que l'on appelle « la plateformisation » du travail. Tous les jours fleurissent de nouveaux services. Il est donc juste de trouver un cadre juridique et social à la hauteur des enjeux, présents et à venir. Notre économie évolue, certes, mais tout comme le marché de l'emploi. Ce n'est pas un secret : les entreprises peinent à recruter. Dans certains secteurs, c'est même dramatique. En première lecture, nous avons déjà évoqué l'hétérogénéité des situations face à l'emploi, la différence entre l'emploi et l'activité, mais aussi la flexibilité que proposent les plateformes numériques, laquelle sous-tend le développement de ces nouvelles pratiques. Ces opportunités économiques correspondent aux évolutions de la société et aux nouvelles habitudes de vie. Cependant, les risques de dérives existent ; ils sont même évidents. Il est donc impératif de créer des mécanismes de protection des travailleurs qui utilisent ces plateformes, qu'ils soient indépendants ou non. Un équilibre reste à trouver. Ce projet de loi a le mérite de nous permettre d'aborder ce sujet majeur pour notre société et de nous interroger sur la meilleure façon de protéger les travailleurs indépendants. Ce sujet est mondial. La Commission européenne a d'ailleurs publié le 9 décembre dernier une proposition de directive pour améliorer les conditions de travail des personnes travaillant une plateforme de travail numérique. Des axes forts y sont défendus sur le droit du travail et la protection sociale. Deux points méritent à mon sens notre attention : le statut professionnel et la transparence sur la gestion des algorithmes. Nous surveillerons les négociations entre les institutions européennes. Il est important d'avoir un cadre européen solide. Quand l'heure de la transposition de la directive sera venue, nous devrons être prêts à discuter de ces sujets. J'espère que, d'ici là, nous aurons mis à profit le temps de la négociation pour entamer une réflexion profonde. Il reste tant à faire pour que l'utilisation de ces plateformes soit synonyme de protection pour les travailleurs indépendants qui y ont recours. au texte lui-même, et je salue le travail effectué par les deux chambres du Parlement. Bien sûr, l'amélioration proposée par le Sénat à l'article 1, qui vise à confier à l'ARPE la mission de réguler le dialogue social entre les travailleurs indépendants et les plateformes de l'ARPE, va dans le bon sens et clarifie le texte.

je regrette le choix de légiférer par voie d'ordonnances. J'aurais préféré que nous débattions plus longuement de ce sujet. Le Parlement a tout de même précisé et encadré certaines parties de l'habilitation. Enfin, la suppression de l'article 3 adopté au Sénat est le signe que nous devons encore approfondir notre réflexion et notre travail. Il est important d'apporter de la flexibilité au cadre que nous souhaitons mettre en place, car il doit pouvoir s'adapter aux évolutions encore nombreuses qui vont se matérialiser. il est important de protéger les travailleurs indépendants en leur permettant d'avoir un dialogue et une relation équilibrés avec les plateformes, afin qu'ils puissent défendre leurs intérêts et obtenir des garanties collectives en fonction des secteurs. Il faut aussi permettre la flexibilité que proposent ces plateformes numériques, tout en l'encadrant sérieusement pour éviter les abus. Le travail qu'il nous reste à accomplir est donc immense, mais les premiers jalons sont posés, cela a été dit à plusieurs reprises. Pour cette raison, le groupe Les Indépendants

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de cette proposition de loi ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées

succédé depuis 2010 ont permis des avancées significatives. Le marché de l'assurance emprunteur pour le crédit immobilier s'est progressivement ouvert à la concurrence. Je rappelle que, avant 2010, chacun devait adhérer au contrat de groupe qui pouvait lui être imposé par sa banque. Les emprunteurs ont depuis lors la possibilité de retenir l'assureur de leur choix, et ce choix n'est plus irrévocable. De plus, la possibilité de résilier son contrat est possible à tout moment jusqu'à douze mois après la signature de l'offre de prêt, puis à chaque échéance annuelle. Ces réformes ont facilité le changement d'emprunteur et ont déjà offert des bénéfices substantiels aux consommateurs. Un bilan des précédentes réformes met en évidence un renforcement de la concurrence et ainsi une baisse de la tarification des contrats d'assurance emprunteur pour le plus grand nombre.

Nous devons toutefois améliorer encore le dynamisme de ce marché et la protection du consommateur, au bénéfice de tous. De nombreux acteurs, dont les associations de consommateurs, se font l'écho de difficultés concrètes rencontrées par nos concitoyens pour substituer le contrat proposé par la banque par un contrat alternatif, au travers d'une délégation d'assurance. La possibilité de changer à tout moment son contrat d'assurance, qui, je le rappelle, fut soutenue par tous à l'Assemblée nationale,

Lors des dernières discussions, le Gouvernement avait rappelé la nécessité de traiter le sujet de la résiliation infra-annuelle de manière consensuelle au sein du CCSF, je regrette qu'aucun consensus de place n'ait émergé. Cette proposition de loi vient à point nommé. Elle est juste et protectrice du pouvoir d'achat des Français, un sujet qui est à l'ordre du jour. Comme nous l'avons fait dans d'autres domaines, nous entendons être au rendez-vous des attentes. Le Gouvernement soutient donc les mesures permettant de rendre le dispositif de résiliation pleinement opérationnel : la transparence des décisions de refus de substitution d'assurance, la meilleure information des assurés, l'introduction d'un délai de production de l'avenant au contrat de crédit lors d'une substitution d'assurance, ou encore le renforcement des sanctions administratives à l'encontre des prêteurs et des assureurs aux pratiques dilatoires. Tout cela permettra de rapprocher le régime

Le Gouvernement veille enfin, tout particulièrement, à l'effectivité de ces réformes menées au bénéfice de nos concitoyens. Il sera nécessaire de prévoir un bilan de la mise en oeuvre de la résiliation infra-annuelle, par exemple un an ou deux ans après l'entrée en vigueur de la mesure.

a pour objet d'élargir l'accès à l'assurance et à l'emprunt des personnes ayant ou ayant eu un problème de santé. Leurs travaux ont permis de grandes avancées en

de santé. La grille de référence Aeras offre également des possibilités plus larges d'accéder à l'assurance de prêts. Ce cadre conventionnel est essentiel pour favoriser l'accès à l'assurance des plus fragiles, afin que les candidats à l'emprunt ne subissent pas une double peine, avec des refus, des exclusions de garanties et des surprimes importantes pour raisons de santé. Il repose non sur l'occultation des situations personnelles, mais sur l'encadrement des pratiques à l'égard des plus fragiles. C'est le seul moyen efficace de garantir que les assureurs continuent d'assurer les plus fragiles dans des conditions raisonnables. À l'inverse, supprimer le questionnaire, comme cela a été proposé à la majorité par la commission,

pour un modèle qui repose sur la protection des plus vulnérables, en encadrant les pratiques et en intégrant tous les acteurs- banques, assureurs, associations -dans une convention de place. La collégialité des décisions relatives à l'évolution de la grille de référence Aeras et au

Madame la présidente, monsieur le ministre,

au sujet de cette proposition de loi, et qui caricaturent inutilement les positions des uns et des autres. Nous entendons souvent, par exemple, que cette proposition de loi permettrait enfin d'ouvrir à la concurrence ce marché, comme si elle allait le faire passer de l'ombre à la lumière, comme si ce marché était aujourd'hui fermé, comme si tout ce qu'avait voté le Sénat jusqu'à présent n'avait jamais existé. c'est tout à fait faux. La concurrence existe déjà sur ce marché, et elle fonctionne bien. J'en veux pour preuve les conclusions du rapport du CCSF de 2020. Tout le monde s'inspire de ce travail, adopté par consensus entre les associations de consommateurs, les assurances et les banques,

la part de contrats alternatifs dans les ventes d'assurance emprunteur progresse régulièrement pour atteindre 25,5 % de la production annuelle ». En trois ans, les contrats alternatifs nés grâce à la concurrence se taillent donc déjà une part de marché de plus d'un quart du flux. Deuxièmement, « les acteurs non bancaires de la délégation/substitution d'assurance- c'est-à-dire les assureurs alternatifs -ont connu une croissance de leur production en nombre de contrats- +46 % pour les assureurs et grossistes et +6 % pour les intermédiaires d'assurance

l'un des effets majeurs des réformes et du développement de la concurrence observé sur le marché, au-delà de la multiplication des acteurs, est la baisse du prix de l'assurance emprunteur. » Au total, la baisse des tarifs a atteint 40 % depuis trois ans. Mes Mes chers collègues, des prix qui sont presque divisés par deux, 50 % de croissance pour les assureurs alternatifs et une part de marché d'un quart des nouveaux contrats : il me semble que nous sommes justement parvenus à instaurer une concurrence vertueuse sur ce marché, et nous pouvons en être fiers, car l'étape clé a

face à cette pression, elles ont créé de nouveaux types de contrats, plus individualisés, notamment pour les profils sans risque. C'est très exactement ce que l'on attend de la concurrence.

Enfin, avant de vous présenter nos travaux, je souhaite revenir sur une autre fausse information qui circule : non, la résiliation à tout moment ne permettra pas de rendre entre 5 000 euros et 15 000 euros aux consommateurs. J'ai dit : « Jusqu'à

du Trésor, qui relève du ministère de l'économie et qui soutient la proposition de loi, estime que le gain est en moyenne de 1 300 euros sur dix ans. Ce n'est pas rien,

quasiment pas d'effet positif, mais qu'elle comporte des risques majeurs que nous devons à tout prix éviter, car le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je le répète, il ne faut pas croire aux économies de centaines de millions d'euros qui sont brandies pour impressionner. Mes chers collègues, j'en conviens, la résiliation à tout moment est un concept qui a l'air séduisant, qui a l'apparence du bon sens, mais nos deux commissions, après des travaux poussés, ont constaté qu'il n'en était en réalité en effet que les avantages de cette mesure sont très faibles. Les assurés peuvent déjà résilier une fois par an, et les profils que cela intéresse l'ont déjà fait. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, le problème ne réside pas dans ce délai de deux mois à respecter.

qui font des économies en résiliant sont souvent des cadres, qui sont au courant de leurs droits et qui n'ont pas besoin de la loi pour savoir qu'ils peuvent partir. Soit vous bénéficiez de la résiliation, et cette loi ne change rien pour vous ; soit vous gagnez en résiliant, et cette loi est donc inutile.

trois ans. C'est peut-être cynique, mais c'est ainsi que cela se passe : les banques anticipent le flux et compensent leurs marges en exigeant des tarifs plus élevés sur tous ceux qui ne peuvent pas jouir de la concurrence, c'est-à-dire les profils au-delà de 45 ans ou de 50 ans, ou les publics fragiles, ou les ouvriers, les employés, etc. etc. C'est cela qui est passé sous silence dans le débat public. Personne n'en parle, alors qu'il s'agit d'un fait majeur. S'il n'y avait pas de concurrence sur le marché, je vous proposerais évidemment de voter la mesure,

! Ces sujets, mes chers collègues, restent de faible importance, au regard des avancées inédites que nous avons actées en commission s'agissant du questionnaire médical. Je suis sûr que nous connaissons tous ici des personnes qui ont été frappées par la maladie qui se sentent empêchées d'élaborer un projet de vie, car on leur refuse l'accès à la propriété, ou alors on le leur consent à des tarifs prohibitifs. Cette situation est injuste et déshumanisante, d'autant plus qu'elle frappe également les personnes guéries. Comment, dès lors, se reconstruire et tourner la page si vous êtes constamment ramené à votre maladie, alors même que vous avez triomphé d'un combat long et douloureux ? Pourquoi exiger des surprimes pour le diabète, pour le cholestérol ou pour le VIH, alors que l'espérance de vie des personnes concernées est la même que pour les autres ? Combien de jeunes sont ainsi empêchés de mener une vie normale, d'accéder à la propriété, de se projeter dans l'avenir ? Nous avons donc supprimé le questionnaire médical pour un grand nombre de prêts immobiliers, dans une logique de justice et d'égalité. J'ai conscience qu'il faut aller encore plus loin et je vous proposerai des amendements en ce sens dans quelques minutes, notamment pour réduire le délai du droit à l'oubli et pour augmenter le plafond de prêt.

avis. Madame la présidente, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, la commission des finances s'est saisie pour avis de cette proposition de loi. J'ai conduit mes travaux en plein accord avec Daniel Gremillet, rapporteur au fond, et nos deux commissions ont adopté des amendements identiques, qui sont désormais intégrés au texte que nous examinons aujourd'hui. Les éléments de la proposition de loi ont déjà été exposés par le rapporteur au fond. Pour ma part, je suis parti du principe selon lequel un système d'assurance a vocation à permettre une solidarité entre assurés et ne doit pas oublier les plus fragiles au profit exclusif de ce que les assureurs appellent les « bons risques C'est pourquoi nous avons proposé une mesure ambitieuse : la suppression du questionnaire médical, afin de permettre aux profils les plus risqués d'accéder à la propriété sans devoir attendre des années pour bénéficier du droit à l'oubli. Le Gouvernement s'oppose, étrangement, à cette suppression, pour des raisons difficiles à comprendre. Le questionnaire de santé conduit, en effet, à appliquer des surprimes, qui n'ont parfois plus de lien avec le risque réel sur l'espérance de vie, compte tenu des progrès médicaux. Dans le dispositif que nous proposons, les prêts concernés seraient remboursés au plus tard à 65 ans, c'est-à-dire à un âge où le risque de décès ou d'invalidité reste encore limité, puisque l'on a encore une vingtaine d'années d'espérance de vie. Les assureurs seront donc donc toujours en mesure de répartir les risques entre les assurés. Le montant des primes pourra être déterminé par d'autres critères que le questionnaire de santé, tels que l'âge, la profession, le montant emprunté ou la localisation du bien acquis. En outre, les données médicales manquent souvent pour donner un fondement objectif aux surprimes. Pour les emprunteurs porteurs du VIH, la surprime appliquée à la garantie décès peut s'élever jusqu'à 100 alors que leur espérance de vie est désormais semblable à celle des personnes non porteuses. Au total, le questionnaire médical s'apparente à un révélateur de risques très perfectible. Il est donc naturel de le supprimer pour la plupart des emprunteurs. Peut-être le montant maximal de 200 000 euros ou le seuil d'âge de 65 ans doivent-ils être discutés ; nous le ferons. Nous devons en débattre, de manière que le Sénat, une nouvelle fois, fasse progresser le système de l'assurance emprunteur au bénéfice de tous, de manière plus volontariste que la simple incitation à négocier qui figurait dans le texte transmis par l'Assemblée nationale. L'autre nécessité est de faciliter l'exercice du droit de résiliation. Disons-le encore, ce droit existe, et la concurrence est déjà réelle sur le marché de l'assurance emprunteur. Un quart des contrats d'assurance emprunteur sont aujourd'hui des contrats alternatifs, grâce aux évolutions législatives survenues depuis dix ans. Le prix de l'assurance emprunteur a baissé pour toutes les catégories, selon le CCSF, sauf, semble-t-il, pour les plus de 55 ans. Ce dernier point doit nous alerter, car, quoi qu'en disent certains acteurs, il existe un vrai danger qu'une généralisation des contrats alternatifs ne conduise à une moindre mutualisation des risques entre assurés. Avec la résiliation à tout moment, on peut craindre que « la péréquation entre " bons risques " et " mauvais risques ", mécanisme naturel dans une assurance, ne se [fasse] plus je cite ici les propos du Gouvernement, représenté par Mme Agnès Pannier-Runacher devant l'Assemblée nationale, le 2 octobre 2020. La position prise aujourd'hui par le Gouvernement

vingt ou vingt-cinq ans. Nous devons nous préoccuper des plus fragiles. Je crains aussi que la résiliation à tout moment n'aboutisse à une multiplication des actions de démarchage, alors même que les démarcheurs en assurance ne suivent pas toujours les bonnes pratiques, comme le rappelle un rapport récent du CCSF.

et connue des emprunteurs, car ceux-ci seront informés chaque année de leur droit de résiliation, comme l'a prévu la commission des affaires économiques. Le texte de la proposition de loi, tel qu'il a été enrichi par l'examen en commission, permettra ainsi de réduire très fortement les risques de manoeuvres dilatoires de la part des prêteurs. Nous avons l'occasion de supprimer les injustices dont certains font l'objet en fonction de leur état de santé et de préserver un bon niveau de mutualisation. Nous sommes contre la dérégulation, monsieur le ministre, et nous sommes favorables à la mutualisation. Tel est mon état d'esprit et la position qui a été prise par la commission des finances. La parole de loi. La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires économiques,

nous examinons la proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur. Ce sujet a été maintes fois abordé ces dernières années, certes, mais il est important pour le pouvoir d'achat des Français et pour tous ceux qui s'engagent dans un contrat de prêt avec une banque.

au Sénat en 2019. Cependant, 87,5 % des contrats d'assurance sont encore détenus par des bancassureurs. Malgré sa libéralisation formelle, le marché de l'assurance emprunteur reste donc, dans les faits, un quasi-monopole bancaire.

de résilier leur contrat quand ils le souhaitaient, de manière à obtenir le taux d'assurance le plus favorable possible. En ce sens, la disposition phare du texte initial, à l'article 1, permettait de répondre en partie à ces problématiques, en ouvrant la possibilité de résilier sans frais et à tout moment les contrats d'assurance emprunteur pour des crédits immobiliers, et en imposant plus de transparence aux banques. Cette mesure bienvenue fut adoptée à l'unanimité à l'Assemblée les modifications adoptées en commission mettent un coup d'arrêt à ce consensus en revenant au dispositif actuel de résiliation annuelle, réduisant quasiment à néant la portée de la

La situation actuelle ne fonctionne donc pas ! Le risque mis en avant par les établissements bancaires quant au danger d'une démutualisation de l'assurance emprunteur nous paraît très largement exagéré : ces contrats sont tous extrêmement rentables, ce qui écarte de fait l'hypothèse que certains risques ne soient plus assurables avec la résiliation à tout moment. La crainte d'une augmentation généralisée des cotisations des assurés à risques n'est pas avérée, dans la mesure où, comme le relève le rapport du CCSF de 2020, les assureurs alternatifs disposent déjà de parts de marché significativement plus importantes auprès de ces publics. C'est pourquoi nous proposerons des amendements visant à restaurer la rédaction issue des débats à l'Assemblée nationale, afin d'obliger les banques à proposer des offres aussi compétitives que les compagnies d'assurances. à cet article 1 totalement dénaturé, nous soutiendrons cependant les mesures qui tendent à renforcer globalement l'information des consommateurs et à lutter contre les manoeuvres dilatoires des banques. En ce sens, nous soutenons l'information annuelle relative au droit au changement d'assurance emprunteur. Nous proposerons également, par amendement, l'augmentation des sanctions administratives en cas de manquement aux obligations de transparence relatives au droit de résiliation. Concernant le second volet du texte, qui tend à faciliter l'accès à l'emprunt et à l'assurance emprunteur des personnes ayant été atteintes de pathologie de longue durée, nous sommes, bien sûr, favorables à toute disposition allant vers une évolution du droit à l'oubli et vers une meilleure prise en compte des personnes atteintes de maladies graves, qui connaissent aujourd'hui de grandes difficultés pour trouver une assurance. Nous souscrivons également à la suppression du questionnaire médical, décidée en commission, car ce document est insuffisamment encadré aujourd'hui. Cela facilitera l'accès à la propriété

En conclusion, si les mesures initiales de ce texte devaient entraîner un transfert de revenus non négligeable des banques vers les emprunteurs et vers les assurances, et participer ainsi à la lutte contre les rentes bancaires, nous regrettons fortement, vous l'aurez compris, mes chers collègues, que le texte issu de la commission y mette un coup d'arrêt.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons un texte qui porte sur l'accès au marché de l'assurance emprunteur. En somme, mes chers collègues, nous débattons pour tenter de rationaliser le capitalisme,

en matière d'assurances emprunteur, les établissements bancaires s'arrogent la part du roi, soit 88 % d'un marché colossal de 7 milliards d'euros. Pour ce faire, ils n'hésitent pas à s'adonner à des entraves à la concurrence par des de clarté des documents précontractuels, des délais prévus au plus court entre la remise des documents et la signature de l'offre, une faible marge sur le crédit au profit de l'assurance pour attirer des emprunteurs ou encore des entraves à la résiliation. Le capitalisme de marché rejette donc la notion même de concurrence, qu'il se plaît à appliquer à tous les autres dès qu'une activité lui échappe. Nous voilà donc face à un paradoxe : doit-on réintroduire du libéralisme afin de prémunir les emprunteurs des pratiques détestables auxquelles se livrent acteurs du secteur ? Avant de répondre, je m'autorise un petit détour historique. L'histoire de la collectivisation des risques individuels est intrinsèquement associée au mutualisme. Elle s'est construite en s'opposant au principe d'une relation contractuelle fondée sur le « chacun paye selon ses risques Au XIX siècle, les sociétés de secours mutuels, avant tout ouvrières, se fondaient sur un lien d'association, une logique d'entraide réciproque qui allait à l'encontre de la logique d'équivalent, le donnant-donnant, propre à l'idéologie marchande. Ce lien concret se manifestait tant dans l'espace public qu'au travail ou dans la sphère privée : veillée des malades et des morts, soins aux veuves ou aux orphelins. L'assurance commerciale était alors rejetée par les milieux populaires. Progressivement, l'entraide et les logiques mutualistes du quotidien ont cependant cédé le pas à la marchandisation et la bureaucratisation, en dissociant l'économique et le social. Aujourd'hui, quel est le niveau de mutualisme et de collectivisation des risques en matière d'assurance emprunteur ? Il est quasiment inexistant. Il a fallu créer une convention Aeras pour forcer gentiment la main aux assureurs en tout genre, afin qu'ils mutualisent les risques ou plutôt qu'ils s'accordent sur des pratiques communes.

Les profils à risques sont donc délaissés par les établissements bancaires qui préfèrent choisir les « bons risques », tout en se délestant de ceux qui leur feraient l'affront de tomber malades ou de l'être Nous proposerons donc un amendement visant à ce que tout individu puisse bénéficier d'un taux fixe pour les garanties décès et invalidité. Je réponds maintenant à ma question initiale sur la libéralisation du marché pour améliorer la concurrence. Il faut faute de mieux, c'est-à-dire à défaut de pouvoir fixer des prix uniques, comme c'était le cas auparavant, selon des critères non intrusifs et objectivables. Faute de mieux, il faudra mettre fin au cartel bancaire en situation de quasi-monopole, qui bénéficie d'avantages disproportionnés et fixe les conditions du marché. Faute de mieux, car des individus se voient encore appliquer des surprimes de plusieurs dizaines de milliers d'euros et doivent pouvoir se libérer du joug de ce vol caractérisé. Faute de mieux, car 68 % des primes reçues ne sont à ce jour pas décaissés. La lucrativité de cette activité n'est plus à démontrer.

la possibilité de supprimer son assurance à tout moment et non plus seulement la première année, puis à date anniversaire. Cette disposition aurait selon nous favorisé favorisé les personnes les moins informées, celles qui n'ont pas négocié avant d'emprunter, celles qui ont subi les prix les plus élevés et les conditions de garantie les plus faibles, celles qui ont eu peur de ne pas pouvoir emprunter, celles enfin qui ne sont pas des fins connaisseurs du secteur

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'achat d'une résidence principale constitue un objectif de vie pour une très grande majorité de Français. En effet, d'après un sondage Harris du mois de décembre 2021, ils sont 76 % à considérer qu'il faut être propriétaire avant la retraite. C'est un objectif stable dans le temps, car il est rassurant, notamment dans la perspective de cette période de retraite. Malgré la crise, cette volonté n'a pas faibli. Elle a simplement évolué et le type de logement recherché a changé : désormais, les Français sont 55 % à privilégier les espaces extérieurs et 52 % la taille du logement. En outre, l'immobilier reste une valeur refuge pour l'investissement. Selon un autre sondage du mois de septembre 2021, les trois quarts des Français aimeraient investir dans le locatif. Ils sont même 11 % à considérer que la crise sanitaire a renforcé leur intérêt pour l'investissement immobilier. Cette situation nous conduit à envisager l'achat immobilier comme étant au coeur des préoccupations quotidiennes des Français. Par conséquent, les conditions d'obtention d'un prêt, notamment les dispositifs d'assurance emprunteur immobilier, doivent nous mobiliser. Le Parlement, en particulier le Sénat, s'est régulièrement intéressé à ce sujet. Depuis dix ans, les conditions d'obtention et d'assurance des prêts immobiliers ont largement évolué. C'était nécessaire.

À chaque fois, les objectifs de ces réformes allaient dans le même sens : améliorer la transparence des processus pour les consommateurs, réduire les coûts d'emprunt en ouvrant le marché, en particulier assurantiel, tout en garantissant la qualité des emprunts et des assurances.

nous manquons de données tout à fait objectives, stables et utilisables pour en juger. C'est d'ailleurs l'une des premières critiques que nous pourrions adresser au secteur de l'assurance emprunteur. que nous examinons la proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur, il ne s'agit pas de distribuer les bons et les mauvais points ni d'avantager les uns ou les autres.

pour les emprunteurs : manque de transparence des dispositifs existants et des décisions des banques, faiblesse de l'information du consommateur, freins dans l'accompagnement des publics les plus fragiles. Sur ces trois axes, nous saluons le travail réalisé par les deux rapporteurs et par la commission saisie au fond pour clarifier la notion de date d'échéance, obliger les banques à informer l'emprunteur de son droit à résiliation annuelle, à justifier complètement les motifs des refus

ces dispositions, même sans la résiliation infra-annuelle, le texte sort renforcé de nos travaux, au profit des consommateurs. C'est pourquoi le groupe Union Centriste votera en faveur de cette proposition de loi, telle qu'elle résulte de l'équilibre trouvé en commission. La parole

Le marché de l'assurance emprunteur concerne des millions de Français, sur tout le territoire. Bien que la souscription d'une assurance ne soit pas juridiquement obligatoire, elle est très courante lors de l'octroi d'un prêt immobilier.

C'est un processus long. Les marges de manoeuvre des emprunteurs se sont significativement accrues ces dernières années, même si le manque d'information des consommateurs sur leurs droits et certaines mauvaises pratiques persistent. de loi que nous examinons s'inscrit dans ce mouvement de renforcement des prérogatives des emprunteurs face aux assureurs. Elle prévoit la possibilité de résilier, non pas une fois par an, mais à tout moment, tout contrat d'assurance emprunteur. Telle qu'elle a été adoptée à la quasi-unanimité par les députés, elle pourrait marquer un renforcement significatif des droits des emprunteurs. Toutefois, le travail accompli par la commission des affaires économiques, la semaine dernière, est venu nuancer ce résultat.

dernière modification, et non des moindres, elle a supprimé, sous certaines conditions, le questionnaire médical. Aussi, je comprends mal la décision du rapporteur de réécrire l'article 1 de la proposition de loi, en le vidant de l'essentiel de sa substance. Le risque de « démutualisation » qu'il invoque ne paraît pas convaincant, puisque les profils jugés à risque se voient déjà appliquer des surprimes et des exclusions de garantie non négligeables.

en rehaussant le plafond de suppression du questionnaire médical pour mieux tenir compte de la réalité des prix de l'immobilier, notamment en région parisienne et dans les grandes agglomérations. Nous voulons enfin renforcer le droit à l'oubli pour les personnes atteintes d'affections comme le cancer ou le VIH, pour lesquelles les restrictions en vigueur n'apparaissent plus forcément justifiées au regard des progrès de la médecine.

Longtemps considérées comme à l'abri de la hausse des prix parisiens, de plus en plus de grandes villes et de périphéries voient le prix du foncier augmenter. Le phénomène s'est accentué depuis les confinements successifs liés à la pandémie. Les différentes mesures prises pour limiter la hausse des loyers et favoriser l'accès à un logement de qualité peinent à porter pleinement leurs fruits. Les territoires ruraux souffrent quant à eux de l'absence de foncier et de la difficile reconquête des centres-villes anciens, dont les logements ne correspondent pas aux standards actuels. Au moment où le pouvoir d'achat s'impose comme un thème majeur de la campagne présidentielle, l'accès au logement et à la propriété à un prix raisonnable doit donc rester l'une de nos priorités.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, souscrire un prêt immobilier est un acte important dans une vie. Il engage l'emprunteur pour de longues années. Afin de garantir le remboursement en cas d'accident de la vie, un contrat d'assurance est alors signé, le plus souvent, avec l'organisme prêteur. Depuis 2014, les emprunteurs peuvent résilier ce premier contrat d'assurance et en choisir un autre, sur le marché, qui viendra en substitution à condition qu'il y ait équivalence de garantie. La loi Hamon du 26 juillet 2014 a permis la résiliation à tout moment, pendant la première année, et l'amendement Bourquin de la loi du 22 février 2017 la permet à chaque date anniversaire du contrat. C'est en nous inscrivant dans ces pas que nous souhaitons compléter les dispositions déjà adoptées par le Parlement. Il s'agit, en effet, d'assurer une meilleure information de l'emprunteur, d'empêcher les mauvaises pratiques de certains organismes prêteurs, enfin de garantir l'accès au crédit de certaines catégories de personnes qui en sont exclues, au prétexte qu'elles ont souffert de pathologies, L'ouverture à la concurrence du marché de l'assurance emprunteur s'est révélée vertueuse. Elle a entraîné une diminution des prix de l'ordre de 40 % au profit des emprunteurs, sans baisse de garanties. La part des contrats dits alternatifs représente désormais 25 % de l'ensemble de ce marché, qui pèse en France près de 10 milliards d'euros et dont le secteur bancaire continue cependant de capter près de 85 %. Notre volonté est d'améliorer l'information des consommateurs. Aujourd'hui encore, certains emprunteurs ignorent parfois jusqu'à l'existence même du droit à résiliation. est par ailleurs nécessaire de faciliter la résiliation en limitant les diverses pratiques dilatoires des prêteurs. Ces pratiques s'opposent, de fait, à la volonté continue du législateur, en dépit des rappels à l'ordre de l'Autorité de contrôle prudentiel

Cette date sera obligatoirement notifiée à l'emprunteur par le prêteur. En second lieu, il est essentiel de mettre fin aux pratiques dilatoires des banques visant à empêcher la résiliation. L'article 2 renforce l'effectivité du droit de résiliation en encadrant strictement les motivations de refus de substitution d'assurance. L'article 4, quant à lui, encadre plus précisément le délai d'émission de l'avenant. Pour que ces nouvelles dispositions soient observées, il importe que le contrôle administratif soit plus effectif et que les sanctions en cas de manquement soient sensiblement plus fortes. Dans le texte que nous examinons, (DGCCRF) et l'ACPR sont chargées d'effectuer ce contrôle et de sanctionner plus fortement les contrevenants, l'amende pouvant aller jusqu'à 15 000 euros par infraction pour une personne morale. Elles auront, en outre, la possibilité de rendre publiques leurs décisions de sanction, ce qui aura sans aucun doute un caractère dissuasif. Il sera bien entendu nécessaire de renforcer les moyens de ces autorités de contrôle, en particulier ceux de la DGCCRF, pour que ces contrôles soient effectifs. Le législateur que nous sommes doit veiller à la réalité de l'application des lois et à l'effectivité du droit. Enfin, l'emprunt s'apparente souvent à un parcours semé d'embûches pour les personnes qui ont souffert ou qui souffrent de

nous proposons que le questionnaire médical soit purement et simplement supprimé pour les prêts immobiliers inférieurs à 500 000 euros, si le signataire à moins de 62 ans. à moins de 62 ans. Ainsi modifiée par notre assemblée, cette proposition de loi rendra effectif le droit à résiliation. Comme l'a indiqué M. le rapporteur, elle constitue surtout une avancée historique qui permettra un accès plus inclusif et plus solidaire à l'emprunt. La parole est

En permettant aux consommateurs de résilier à tout moment leur assurance emprunteur, sur le modèle de ce qui est déjà possible pour les assurances habitation et les assurances automobile ou moto.

Ce n'est pas rien. Ce texte a donc fait l'unanimité. Aucun groupe politique n'a manqué à l'appel. Pourquoi un tel consensus politique à l'époque, parce que nous sommes nombreux à considérer ce marché comme peu dynamique, très rentable pour les banques et, au contraire, peu favorable aux consommateurs ? Et puis, patatras, machine arrière toute ! la majorité sénatoriale est revenue sur cette belle avancée pour s'en tenir à une information annuelle sur le droit de résilier ces contrats, ce qui existe déjà. Pourquoi ? Officiellement, selon le rapport de M. Gremillet, parce que « la concurrence sur le marché de l'assurance emprunteur fonctionne de façon satisfaisante ». Pardonnez-moi, monsieur le rapporteur, mais lorsque l'on sait que ce marché est détenu à 88 % par les banques ... Cela ne veut rien dire ! ... et à 12 % par les assurances alternatives, j'aurais plutôt tendance à parler de « monopole bancaire réformes qui se sont succédé depuis la loi Lagarde pour libéraliser le marché n'ont pas eu l'effet escompté. En 2019, selon le rapport du CCSF, les banques ont encore réussi à gagner 9 % de parts de marché, avec 136 000 souscriptions de plus qu'en 2018. Dans les faits, les textes ont tenté de resserrer l'étau pour faciliter la vie des emprunteurs. Toutefois, comme nous pouvons le constater dans notre propre vécu ou autour de nous, les mesures dilatoires existent toujours. Par exemple, nous avons le droit de changer d'assurance à date d'échéance, mais cette date, qui la connaît hormis la banque ? Deuxième argument avancé, la résiliation infra-annuelle (RIA) pénaliserait surtout les personnes les plus fragiles.

termes, comment le fait de pouvoir choisir librement à tout moment sa date de résiliation pourrait mettre en difficulté les personnes les plus fragiles ? J'avoue tourner le problème dans tous les sens, je ne comprends pas. Je veux revenir, par ailleurs, sur la suppression du questionnaire de santé, acté par un autre amendement phare du rapporteur. Le sujet n'est pas simple. Il paraît difficile d'accepter qu'il puisse exister encore des discriminations sur des critères de santé dans le domaine des assurances. L'article 7 de la proposition prévoyait que les signataires de la convention Aeras engagent rapidement une négociation afin non seulement de réduire les délais du droit à l'oubli pour les pathologies cancéreuses, mais aussi d'étendre la grille de référence Aeras à d'autres pathologies ou maladies chroniques.

D'une part, les assureurs n'auront pas d'autres choix que de prendre ce risque sur leur portefeuille et de le mutualiser par une prime de risque qu'ils feront partager à tous les assurés,

Malgré le beau message que constitue la suppression du questionnaire médical, le diable se cache dans les détails. Oh là là ! Une telle mesure doit faire l'objet de discussions sérieuses, avec tous les acteurs concernés. la commission des finances, en séance, lors de l'examen du dernier projet de loi de finances, « pour atteindre les objectifs que l'on se fixe en la matière, il ne suffit pas de claquer des doigts et de le demander : il faut regarder de manière plus approfondie quelles contraintes s'imposent Mes chers collègues, nous avions dans les mains une belle proposition de loi, nous avons désormais un objet politique clivant, au détriment des consommateurs. Nous regrettons le choix qui a été fait par la majorité sénatoriale. Par nos amendements de rétablissement, nous essaierons de vous faire entendre raison. Dans le cas contraire, nous faisons confiance à la navette parlementaire pour décadenasser définitivement ce marché, dans l'intérêt des emprunteurs. La

la France a beau être la patrie de Tocqueville, la liberté individuelle pâtit chez nous d'une image à tout le moins mitigée. Le mot reste attaché à un imaginaire sauvage, où David doit affronter Goliath sans sa fronde.

c'est tout l'inverse, monsieur le ministre. La libre concurrence, en particulier, a pour vocation première d'établir des règles qui garantiront la liberté de chacun, singulièrement la liberté des faibles contre la liberté des forts. L'ambition du libéralisme économique, c'est que cette organisation, fondée sur des règles et sur la liberté, contribue à rendre notre société tout à la fois plus prospère, plus tolérante et plus juste. cette proposition de loi nous offre un cas d'étude intéressant. Elle vise spécifiquement le marché de l'assurance emprunteur et elle y introduit davantage de liberté, en permettant à l'assuré de résilier son contrat à tout moment. L'enjeu est important, car ce changement des règles du jeu devrait générer de nouvelles opportunités économiques, en introduisant la concurrence là où les acteurs établis disposent d'une position de force qui ressemble fort à une rente.

Je me contenterai de revenir sur trois arguments avancés par les rapporteurs contre cette mesure. Le premier argument porte sur la compétitivité présumée des offres d'assurance crédit sur le marché, Daniel Gremillet. On nous explique que, si les banques détiennent encore 88 % des parts de marché- j'ai noté que nous n'étions pas d'accord sur le chiffre -, c'est non parce qu'elles font de la rétention de clientèle, mais parce qu'elles proposent des offres très compétitives pour les assurés.

Mieux vaut encadrer les pratiques que de supprimer les offres qui peuvent donner lieu à un démarchage- ou alors, il faudrait tout bonnement administrer toute l'économie, mais je ne crois pas que cela reflète la volonté de la majorité. Le troisième argument porte sur la déstructuration du marché et la liquéfaction complète de la demande, qui rendraient toute offre solide En permettant aux emprunteurs de résilier leur contrat quand ils le souhaitent, ils en changeraient tout le temps, comme on zappe devant sa télévision ou comme on déroule un fil d'actualité sur son téléphone. Cette crainte ne correspond pas à la réalité. Les consommateurs n'ont aucune envie de changer sans cesse d'assurance. Ils ont mieux à faire.

Mes chers collègues, je crois que notre rôle est de défendre le faible plutôt que le fort, en l'espèce le consommateur plutôt que la banque ou l'assureur. Je vous proposerai des amendements en ce sens. Nos rapporteurs ne s'y sont d'ailleurs pas totalement trompés, puisqu'ils ont proposé une mesure importante sur la suppression, sous certaines conditions, du questionnaire de santé pour l'établissement d'un contrat d'assurance emprunteur.

que les assurances proposent des offres dégradées aux personnes qui ont vaincu un cancer ou qui souffrent d'une pathologie chronique. De telles discriminations pour raisons de santé

Marqués par la crise sanitaire et les confinements successifs, de nombreux Français, en particulier ceux des métropoles, ont déménagé- ou voudraient le faire -vers des villes à taille humaine, près des littoraux ou à la campagne. Pour les investisseurs, la pierre reste un placement intéressant. Ces démarches vers l'accession à la propriété, qui passent en général par l'obtention d'un prêt, sont, pour certains, ardues et inégalitaires. Bien évidemment, la question des revenus des emprunteurs entre en jeu. Malgré « l'argent à bas coût », on constate un resserrement de l'accès au crédit pour certains profils, comme les plus jeunes ou les plus modestes, qui, en outre, ne disposent pas d'un apport personnel suffisant. De fait, l'application du ratio maximal d'endettement, qui inclut l'assurance emprunteur, augmente parfois significativement la mensualité et conduit au refus de certains prêts. Pour ceux qui obtiennent leur prêt, le prix de l'assurance est une charge pouvant se révéler non négligeable, alors même que l'assurance n'est juridiquement pas obligatoire. Contrairement à un sentiment trop répandu, la question du coût de l'assurance emprunteur n'est pas marginale. Il en va de même pour le choix de l'assureur, puisqu'il est possible de souscrire une assurance emprunteur autre que celle que sa banque Dans les faits, malgré l'accroissement du nombre de contrats alternatifs dans la période récente, les banques dominent encore largement le secteur assurantiel pour les crédits immobiliers. Pressé de vouloir conclure, devant respecter différents délais, l'emprunteur va généralement au plus simple et au plus rapide : l'assurance proposée par sa banque. En ces périodes de taux bas, peu rentables pour les banques, il me semble que l'assurance emprunteur offre à ces dernières des marges confortables. De plus, tous les emprunteurs ne se trouvent pas sur un pied d'égalité. Ceux qui parviennent à faire appliquer leur droit de mise en concurrence sont souvent des cadres les ménages les moins aisés, soucieux d'obtenir leur crédit ainsi qu'un taux attractif, peuvent être contraints d'accepter l'offre d'assurance de la banque. diverses manoeuvres, parfois qualifiées de dilatoires et souvent dénoncées par les associations de consommateurs, rendent les changements de contrat compliqués pour les emprunteurs.

Paradoxalement, compte tenu des différentes contraintes qui leur sont appliquées, en particulier d'importantes surprimes, les personnes à risque en matière de santé sont tout à fait rentables : ce sont d'excellents clients pour les assurances. À raison, les associations de patients, qui mènent un travail remarquable en faveur des droits des malades et des anciens malades, attendent des évolutions, notamment en matière du raccourcissement du délai d'accès au droit à l'oubli de son extension aux pathologies chroniques. En conclusion, il ne s'agit pas de faire des banques et des assurances des boucs émissaires. Très bien ! Elles permettent à de nombreux Français de réaliser leurs projets. Toutefois, il est nécessaire d'aller vers davantage de transparence, d'information et de liberté en faveur du consommateur.

C'est le principe même de la mutualisation qui se trouve mis en cause au profit d'une individualisation des contrats, alors même que le ratio de sinistres à primes reste largement favorable aux assureurs.

en France, l'assurance emprunteur n'est pas obligatoire. Cependant, à la différence de bien des pays, le prêteur l'exige pour se prémunir du risque, notamment en cas de prêt immobilier. Malgré son coût, l'assurance emprunteur a le mérite d'éviter le recours à l'hypothèque, à la caution, au nantissement ou au privilège de prêteur de deniers, ce qui, convenons-en, facilite les transactions. Nous avons$ pris connaissance du bilan détaillé du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) demandé par Bruno Le Maire au mois de juillet 2019. Sur l'ensemble des contrats d'assurance emprunteur, 75 % sont des offres bancaires, 13 % des offres internes aux banques et 12 % de véritables contrats alternatifs. La question se pose : 12 %, est-ce trop ou trop peu ? Quel est le degré de marge sur ces contrats ? Peut-on croire que, sur 100 euros de primes collectées, 32 euros seulement seraient reversés aux assurés, soit une marge deux fois plus élevée que sur les contrats d'habitation et trois fois plus que sur les contrats automobiles ? il s'agit de veiller à la fois à la qualité et à la quantité de l'offre auprès de l'emprunteur. Celui-ci, soulagé d'avoir conclu un accord sur le nominal de son emprunt, n'a bien souvent ni le temps ni l'énergie de batailler sur l'assurance emprunteur, d'où les déconvenues et l'opportunité de la mise en concurrence. La concurrence a produit ses effets. Dans son rapport, le CCSF relève une baisse généralisée des tarifs de 10 % à 40 % selon les cibles et pointe la segmentation tarifaire des contrats alternatifs, faisant craindre une démutualisation du marché. Pourtant, les banques baissent le prix de l'assurance des jeunes emprunteurs, mais relèvent celui des seniors

Il y a donc bien un risque de démutualisation, mais celui-ci se vérifie davantage auprès des banques afin de lutter contre la concurrence et de préserver leur marge. Dès lors, notre marge de progression est réelle. À cet égard, il nous paraît beaucoup plus utile d'apporter davantage de transparence et de lisibilité sur les différentes offres plutôt que de permettre de modifier le contrat à tout moment.

Au moment de souscrire un contrat d'assurance ou d'emprunt, les malades de cancers et d'hépatite C n'auront plus à le mentionner dès cinq ans après leur rémission (contre dix ans aujourd'hui). Nous l'étendrons aussi à de nouvelles maladies. »

Cette convention ne concerne en effet aujourd'hui que les personnes atteintes ou guéries de cancer. La simple négociation prévue dans la version du texte issue de l'Assemblée nationale n'est pas satisfaisante. Nous estimons qu'il faut inscrire cette extension aux autres maladies chroniques

Notre objectif est simple : il vise à rendre la convention Aeras plus inclusive, plus facile d'accès et plus efficace pour toutes les personnes atteintes de pathologies chroniques ou de cancers. Quel dommage

Pourtant, dans cet hémicycle, je dois être l'une des rares parlementaires à avoir participé activement aux débats des lois Chatel, Lagarde, Hamon et de l'amendement Bourquin. J'ai même travaillé avec ce dernier sur les dispositions votées dans la loi C'est dire si je mesure le chemin parcouru en une décennie sur les modalités de résiliation de cette assurance, qui a toujours été à part. J'étais donc persuadée que les dispositions de 2020 étaient effectives. Rappelons qu'elles avaient fait l'objet de concertations avec différents intervenants et qu'elles clarifiaient le droit à changer d'assureur après un achat immobilier- une possibilité acquise très progressivement grâce aux nombreux combats menés par les associations de consommateurs et par les parlementaires. Reconnaissons que le juste milieu entre la protection du consommateur, l'équilibre financier indispensable aux assureurs et l'ouverture du marché aux intervenants alternatifs n'est pas forcément facile à trouver.

je me réjouis des travaux menés par le rapporteur Daniel Gremillet et les membres de la commission des affaires économiques : l'adoption de deux amendements, ils ont rétabli la procédure actuelle, autorisant ainsi la démarche de résiliation et de substitution dans les deux mois qui précèdent la date d'échéance du contrat.

la faculté de changer d'assurance emprunteur. Ils réussissent plus facilement à l'imposer à leurs banques, celles-là mêmes qui ont récemment annoncé des profits record pour l'année 2021. À l'heure où le pouvoir d'achat est la priorité numéro un des Français, il n'y a pas de petit gain.

qu'il ne fallait pas laisser croire que les sénateurs, ceux de la majorité en particulier, étaient les porte-parole des banques, quand bien même

aux faibles, c'est-à-dire aux emprunteurs. Ce choix doit se faire en conscience, librement, sans subir d'anathème.

puisque le code de la consommation prévoit déjà que le coût de l'assurance emprunteur doit être mentionné sur tout document fourni à l'emprunteur avant l'offre de prêt qui traite de ce sujet. L. 313-8 dudit code précise que ce coût est exprimé en taux annuel effectif de l'assurance, qui permet la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit.

Il est ainsi proposé que la liste des informations devant figurer dans l'offre de prêt soit complétée par les éléments relatifs aux garanties exigées par la banque pour l'octroi et le maintien du crédit. Cette information est importante, car la banque ne peut pas refuser un autre contrat d'assurance emprunteur s'il présente un niveau de garantie équivalent au contrat initial. Aussi, cette information figurant dans l'offre de prêt prend un caractère contractuel. Non seulement elle permet à l'emprunteur de disposer d'un document de référence

M. Daniel Salmon. La proposition de loi renforce les sanctions administratives en cas de manquement aux obligations de transparence relatives au droit de résiliation. Nous soutenons bien évidemment avec une sanction ne pouvant excéder 3 000 euros pour une personne physique, comme le prévoit actuellement le texte, il reste très rentable pour les banques et autres sociétés financières de ne pas informer leurs clients de la possibilité de résilier leur contrat d'assurance emprunteur. Afin de rendre la sanction réellement dissuasive, il est donc proposé de porter son montant à 12 000 euros pour les particuliers. Afin de conserver l'écart prévu par le texte, ce même montant serait fixé à 60 000 euros pour une personne morale.

Or il semble de bon sens, puisqu'il prévoit que le coût de l'assurance emprunteur soit affiché, non seulement sur la durée du prêt, mais aussi sur huit ans, c'est-à-dire la durée moyenne d'un prêt dans les faits. Ainsi, l'emprunteur pourrait comparer avec plus d'efficacité